la séance et reprise, madame la ministre, mais chers collègues. Par lettre en date du 7 décembre le gouvernement a demandé d'inscrire à l'heure du jour, du lundi 18 décembre après-midi l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire. Sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2017 717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense de compléter l'ordre du jour du mercredi 20 décembre après-midi par l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2017 644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des hordes des professions de santé. Donc acte et donner de ces demandes. Nous pourrions fixer l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2017 717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense le 18 décembre à 15 heures. Et nous pourrions prévoir pour chacun de ces textes une discussion générale de 45 minutes. Qu'il y a des observations sur ces annonces et ces communications. Pas d'observation, donc il en est ainsi décidé. Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi de finances adoptées par l'Assemblée nationale pour 2018, nous sommes parvenus dans l'examen des articles non rattachés à l'amendement numéro 691 rectifier bis au sein de l'article 39 sixties. Donc, c'est l'article 39 sexy, j'ai 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Donc, le 691 n'est pas soutenu, c'était Monsieur Adnot. Le 528 donc, au nom de la commission des finances, Monsieur de Mongolfier.

il y a des différences de traitement qui pouvait se justifier un moment on a voulu aider ce qu'on appelait les mutations de aujourd'hui ces différences de traitement conduit à fragiliser les fonds et je me réfère en terme d'efficacité au référé de la Cour des comptes de 2016 sur l'ISF-PME qui considérait que l'investissement sous forme intermédiaire était sans doute la plus efficace, alors quel est le coût de cette mesure parce qu'on va peut-être nous objecter que cette mesure a un coût, si c'était le cas, on aurait aimé savoir ça fait environ 10 15 jours qu'on a écrit pour avoir des précisions de chiffrage, on les a pas eu donc nous considérons que cette question devait pas être pertinente et que le coût devrait être extrêmement limité et c'est la raison pour laquelle j'habite le Sénat à soutenir cet amendement de la commission des finances. Alors amendements identiques, l'amendement 705 rectifier madame Lamure Madame le Khomeiny. Pour poursuivent l'encouragement à l'investissement des particuliers dans le dans les PME et la délégation aux entreprises recommandent en compensation d'élargir le recours à la réduction hier PME elle préconise notamment que ce dispositif s'applique de manière identique à tout investissement qu'il soit opéré de manière directe ou intermédiaires aujourd'hui, le plafond de versements ouvrant droit à réduction d'impôt est 4 fois plus bas pour l'investissement intermédiaires que pour l'investissement Direct, alors même qu'est ce qu'il est avéré que la performance de ses investissements et souvent meilleure que celle des investissements Directs, la Cour des comptes juge d'ailleurs peut justifier ce traitement fiscal différencié cet amendement propose donc d'unifier le plafond des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sans distinguer entre versements Directs et versement intermédiaire il aligne ces plafonds en relevant les plafonds applicables aux investissements intermédiaire au niveau des plafonds applicables aux investissements Directs. Merci donc l'avis du gouvernement sur ces 2 amendements identiques ni Nice. Merci monsieur le président, monsieur le rapporteur général, mesdames et messieurs les sénateurs. Le calibrage de dispositif Madelin en fonction des modalités d'investissements Directs ou indirects, via des fonds garantis une adéquation entre le risque supporté par le souscripteur et l'Avantage fiscal accordé dans le cas d'un investissement via un fonds l'investissement se répartit sur un grand nombre de PME différentes, ce qui permet de limiter le risque pris par l'investisseur ensuite la réduction d'impôt sur le revenu, Madelin est déjà très favorable et vos proches et vos propositions paraissent excessives, notamment au regard de leur coût pour les finances publiques a été qui est difficile et à évaluer puisqu'il est, il va dépendre des changements de comportement des investisseurs, mais qui a été chiffré entre 10 et 50 millions d'euros. Merci.

quand on est dans une Holding, que je sache, c'est la même situation, une Holding on a par définition des participations qui sont répartis sur plusieurs sociétés, donc c'est ce point de vue assez incohérent et donc c'est la raison pour laquelle aussi au sureau souhaite mette fin à cette incohérence qu'il y a un moment pu justifier et qui, aujourd'hui, les plus pertinentes. Merci donc, s'il n'y a pas d'explication demande d'explications de vote, je vais mettre aux voit ces 2 amendements identiques qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient donc ces amendements sont adoptés, j'ai ensuite en discussion commune 3 amendements

C'est un amendement auquel j'espère grandement poète être favorable puisque il vise tout simplement à ce que l'investissement aille aux entreprises et n'aille pas aux intermédiaires. Tout simplement en plafonnant les frais qui sont perçus par les différents intermédiaires vous souvenez que, à l'initiative de notre commission, nous avions plafonner les frais relatifs à l'ISF-PME toutes les études montrent que c'était efficace conduit à réduire les frais et faire en sorte que l'investissement aille directement dans les autres pays, c'est bien le but on a eu des débats d'ailleurs ce matin concernant l'immobilier locatif aidés du type Pinel dans ce même esprit, nous proposons concrètement comme le fait en 2015 de mettre fin, pratiquer veut puisqu'on voit que les frais perçus par les intermédiaires étaient parfois très élevés par 4,8 pourcent par an en moyenne pour les fonds fiscaux, contre 2 devrait et 5 pourcent pour les faux professionnels et, parfois, parfois,

et grâce à ces justement ça permettra tout simplement que le niveau de frais soient raisonnables sera d'ailleurs a fixé par voie réglementaire et que l'argent investi par les contribuables, en contrepartie d'un Avantage fiscal, c'est vrai, hé bien bénéficie aux entreprises et donc je pense que Allemands pour être favorable,

Oui, c'est un amendement identique de la commission des à de la délégation aux entreprises, donc qui va dans le même sens et parfaitement défendu par notre rapporteur. Très bien, donc l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, merci Monsieur le Président, je, je confirme que nous ne pouvons 4 d'accord avec l'objectif. le les fonds de ce dispositif aillent en priorité aux PME et donc ce plafonnement des frais en cohérence aussi avec ce qui avait été fait sur le dispositif Pinel et c'est une bonne chose, donc nous sommes favorables. Très bien, donc ces 2 amendements avec avis favorable de la commission favorable du gouvernement, je mise aux voix. Pour.

sur cet article qui est pour. Compte. Donc, l'article est adopté article additionnel après l'article 39 sexy.

Donc, le 530 présenté par Monsieur de Mongolfier au nom de la commission des finances, monsieur le rapporteur général. Cet amendement vise à mettre fin à un certain abus ou du moins contournement. D'un dispositif anti-abus qui avait été d'ailleurs votée à l'initiative de la commission des finances, initiative du Sénat puisque nous avions dans la loi de finances rectificative pour 2015

éligibles aux activités au bénéfice des réductions d'impôt ISF et Madelin puisque vous comme vous savez, ces autobus solidaire ne sont pas, par définition, concernés par l'exclusion des activités, donc c'est une forme de contournement de la loi, ce qui était finalement important c'est moins le statut de l'entreprise que la finalité de l'investissement, si c'est une activité de promotion pure que l'entreprise soit une forme de S. d'entreprise solidaire ou telle ou telle forme juridique, c'est finalement peu important, ce qui est important, c'est la finalité : où va la seulement et quelle est la prise de risque, elle est sans doute différente sur la promotion immobilière et donc nous souhaitons mettre fin à ce contournement et gelé les activités trop monsieur, mais vous dire, à l'exception, seulement, bien sûr, de celles relevant du d'une vocation sociale donc, sous cette réserve je vous rappelle qu'il y a également une condition analogue qui existe en matière d'impôt sur la fortune, mais là, nous parlons bien du match. Merci donc sur cet amendement de la commission, l'avis du gouvernement avait ministre. Merci monsieur le président, les us bénéficie de plusieurs conditions dérogatoires dérogatoire dans le cas de cette réduction d'impôt Madelin ce qui atteste de la prise en compte par le législateur des spécificités des entreprises d'économie sociale et solidaire, il est clair qu'en contrepartie de ses décorations de dérogation, il convient de veiller à prévenir tout abus et je partage de ce point de vue, la préoccupation de la Commission, ceci dit. Les services de la DG Philippe non pas à ma connaissance, été alertés de pratiques abusives dans ces conditions, j'ai un avis défavorable à l'amendement et je m'engage auprès de votre assemblée a demandé à mes services d'expertiser plus avant cette question.

Donc, l'amendement est maintenu, il y a pas d'explication de vote je le mets au voix qui est favorable à l'amendement avec un avis défavorable du gouvernement. Comptes.

merci Monsieur le Président, qui ont un modèle économique plus faiblement rentable que les autres attirent peu d'épargne privée et cet amendement propose donc de sortir l'actionnariat solidaire du plafonnement des avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu qui sont prévues à l'article 200 0 A du code général des impôts, merci. Merci donc sur cet amendement, l'avis de la commission. tout à une discussion a Commission européenne qui nous a obligés à réformer le dispositif d'ISF PME sur le Madelin très concrètement le difficile actuelle je vais très directe n'a jamais été notifiée et il faudrait vérifier sa conformité aux règles européennes par rapport aux aides d'État

Donc, il est pour cet amendement. Est content. Qui s'abstient donc l'amendement n'est pas adopté. Alors après, toujours l'article 39 sexy le 707 donc ça doit être madame de Khomeiny. Oui, merci Monsieur le Président, à nouveau, un amendement de la délégation aux entreprises, la suppression de l'ISF-PME doit conduire à rechercher d'autres moyens de soutenir l'investissement dans les PME, un moyen et d'améliorer les dispositifs existants comme le dispositif Madelin hier PME mais aussi comme le compte PME Innovation, créé il y a un an, le compte PME une ovation a été initiée début 2016 par monsieur Macron, alors ministre de l'économie, les personnes physiques impliquées dans la gestion de leur entreprise à réinvestir dans la nouvelle PME les plus-values tirées de la cession de titres de leur société et accompagner le développement de ces PME en les faisant bénéficier de leur expérience et de leur réseau, cette incitation repose sur le report de la taxation à l'hier de ces plus-values jusqu'au moment où les liquidités lié aux plus-values sont retirés du compte PME Innovation lequel fonctionne comme comme un PEA avec compartiment destiné au titre et compartiments destinés aux liquidités en attente de réinvestissement les conditions fixées par la loi de finances rectificative de 2016 pour bénéficier de ce report d'imposition était jugée trop restrictive par la commission des finances du Sénat qui avait bien tenté d'améliorer le dispositif, sans être suivi par l'ancienne assemblée la délégation aux entreprises avaient déploré l'inadaptation du compte PME Innovation dans son rapport de février 2017 appelant à moderniser la transmission d'entreprises en France, en effet, le compte PMU une ovation et moins avantageux sur certains aspects, que le régime de report d'imposition prévue à l'article 150 du code général des impôts en cas d'apport cession de titrent ainsi permet uniquement de décaler l'imposition à l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux qui pourraient s'élever à 17,2 pourcent en janvier 2018, du fait de la hausse de la CSG restant dues au titre de l'année, de réalisation des plus-values dans le Comte, alors que le régime prévue à l'article 150 irait 0 BPR permet également de différer le paiement des prélèvements sociaux, d'après les informations recueillies par la délégation le compte PME Innovation fait effectivement peu d'adeptes, cet amendement propose donc de prévoir aussi le rapport des prélèvements de report des prélèvements fiscaux pour lever l'un des premiers obstacles au succès du compte PME Innovation et encourager ainsi la veste seulement dans les PME parler Business un job. Merci donc sur cet amendement, l'avis de la commission. créé par la finance rectificatif pour 2016, donc il y a peut-être un peu tôt pour en tirer le bilan complet, mais il semblerait que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas très bien, et sans doute l'une des faiblesses du dispositif et celle qui est soulignée par l'amendement, a la possibilité de reporter le devoir d'un différé de paiement pour les prélèvements sociaux, alors peut-être que l'amendement remet dirait remet une de ses difficultés, mais peut-être avant de se prononcer définitivement, je souhaiterais savoir si le gouvernement à la fois un 1er bilan du dispositif et un chiffrage de la mesure qui nous est proposé, qui pourrait être en effet relativement modeste est-ce que ça permettrait en tout cas, d'améliorer l'attractivité du compte PME Innovation qui visait à remédier à ces difficultés de financement des PME. Madame la ministre du gouvernement. du nombre de compte PME Innovation qui qui disent être un peu limité pour effectuer un chiffrage fiables, alors si on peut comprendre l'objectif de cet amendement qui, en effet, le rend plus attractifs et de et et d'inciter à ses investissements dans des dans nous considérons que, à ce stade se compléter, dispositif n'est n'est pas opportun et que ça introduirait un un mécanisme complexe d'étalement et difficile si le nous rappelons que dans le cadre de cette loi de finance de nombreuses très visible avancées ont été faites sur la fiscalité du capital qui nous semble, avec la suppression de l'Yacef et l'instauration du prélèvement forfaitaire unique vraiment répondre à cet objectif d'orientation du capital, donc nous suggérons le retrait de l'amendement. Bien Bien vous retirer l'amendement non, non, l'amendement est maintenu, donc je vais le mettre aux voix avec un avis qui était de sagesse qui était d'attente de la commission et un avis défavorable du du gouvernement qui est favorable à cet amendement. Qui est contre. L'amendement est adopté. dont 8 rectifier toujours madame de Khomeiny. Oui, Monsieur le Président, poursuivant son objectif d'instaurer un véritable dispositif de compte entrepreneur investisseur permettant aux dirigeants d'entreprises, de soutenir plus activement la croissance des PME françaises, la délégation aux entreprises juge indispensable d'assouplir le recours au compte PME Innovation pour assurer le succès cet amendement propose de revenir sur 2 contraintes particulièrement pénalisante qui contribue au manque d'engouement pour ce dispositif censé favoriser le développement de l'écosystème français des Business, il il propose de ramener de 25 pourcent à 10 pourcent la part des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux dont la détention est requise dans les sociétés dont le titulaire de ces pays souhaite déposer départ sur le CPI il rationalise les conditions d'accompagnement prévues en cas d'investissement intermédiaires dans les PME via un fonds en effet les investisseurs doivent fournir leur expertise aux PME qu'le finance et pour cela, signer avec elle une convention d'accompagnement prévoyant leur participation à l'élaboration de la stratégie de ces PME et la fourniture de conseils à titre gratuit s'il investit s'il investit non pas directement dans les PME, mais via un fonds chacun des investisseurs titulaire d'un CPI doit signer une telle convention avec chacune des PME dans lesquels ce fonds investi ce qui est d'une grande lourdeur la amende l'amendement propose de simplifier les choses, en prévoyant que la convention soit mise en place au niveau du fond et non de chaque investisseur individuel.

qui n'avait malheureusement pas été repris ensuite par l'Assemblée, donc, évidemment, pour les mêmes raisons que Lerner c'est la commission et emporté ces dispositions sur le le père le compte PMU innovation il y a, par définition très favorable. Merci la vie du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, merci Monsieur le Président, donc à nouveau ce ce dispositif et est très récent, nous n'avons pas d'évaluation, et nous avons comme vous le savez, un travail en cours de discussion sur le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises qui doit aborder en particulier tous les obstacles à leur financement s'agissant bien évidemment aussi des des PME, donc je pensé plutôt dans le cadre de de ce de ce plan que nous souhaitons revenir sur ce sujet et discuter avec les acteurs de leurs attentes, donc avis défavorable sur cet amendement. Pas d'explication de vote donc je mets aux voix cet amendement avec un avis favorable de la commission NAVY défavorable du gouvernement. C'est pour.

Qui est contre. Abstention donc cet article est adopté. Ensuite, après cet article 39 cèpes. Teaser donc article additionnel. J'ai un amendement de alors monsieur ou Madame Dumas, pardon, j'ai pas vu. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, alors il s'agit d'un amendement qui concerne le cinéma français, son rayonnement qui tient pour bonne partie à la qualité de la production des premiers et deuxièmes films ainsi que des films à faible budget l'offre cinématographique doit participer non seulement au renouvellement et à la diversité de la création, mais également à l'émergence de jeunes talents, qu'ils soient, réalisateurs, acteurs ou techniciens mais sans le soutien, ou avec un soutien marginale des investisseurs privés, ces réalisateurs émergents sont souvent soutenus par des mécanismes très sélectif de financement public, comme l'avance sur recettes, les aides régionales et il ne peut bénéficier du crédit d'impôt pour les dépenses de production déléguée en effet la part de financement public dans les films à petit budget et proportionnellement plus importante, ce qui les contraint à renoncer au crédit d'impôt pour respecter le plafond de 60 pourcent du budget de production, et c'est là le problème, ce présent amendement qui a été déjà proposé par la députée de Paris, Brigitte Kuster, à l'Assemblée vise à porter ce seuil à 70 pourcent afin de leur assurer un accès effectif au crédit d'impôt et garantir une égalité des films face à ce dispositif, un article d'un grand quotidien paru lundi dernier, après le vote à l'Assemblée, décrit parfaitement la situation et souligne que la législation française est la plus dure d'Europe, la ministre de la culture, d'ailleurs, affirmait encore récemment qu'il n'y a jamais de trop de création et que ce dynamisme est une force dans un monde ouvert plus de 2000, scénaristes, réalisateurs, producteurs viennent d'ailleurs de faire une pétition et porté notamment par les plus grands noms dans ce sens, donc, l'occasion est donc donnée à la ministre de la culture d'assurer une plus grande égalité entre les films face au crédit d'impôt.

assez puissants, qui d'ailleurs se soit félicité a permis en France contrairement à beaucoup de pays d'Europe, le maintien d'un cinéma français, donc il y a une industrie cynotechnique en en France, et c'est là peut-être dû au talent et sans doute, mais également due un ensemble de dispositifs fiscaux, budgétaires extra-budgétaires 2 de soutien d'avances sur recettes etc qui permet de soutenir la production c'est le de graphiques

plus les plus élevés, et donc en augmentant de de 60 pourcent à 70 pourcent la part des financements publics et peuvent recevoir les films difficiles à petit budget, on irait sans doute encore plus loin et ne paraît pas à ce stade opportun de relever encore ce plafond, dans les amendements suivants va voir dispositif sur le théâtre, le théâtre, vous verrez, malheureusement il a pas de dispositif aussi puissant et secret en avoir, je pense qu'il faut rester en équilibre par rapport à jeudi à à discuter de soutien au cinéma qui ne se limite pas simplement ce dispositif mais qui, je le rappelais bénéficier à la fois de financement budgétaire extra-budgétaires et fiscaux. Merci vie du gouvernement mais Oui, merci Monsieur le Président, en effet, les dispositifs de soutien sont sont puissants sont nombreuses secret des impôts a été très largement renforcé ces dernières années, le taux de subventionnement et est très élevé, donc nous sommes défavorable à l'amendement.

Merci monsieur le président, monsieur le rapporteur général, Madame la Ministre, juste moi je souhaite soutenir cet amendement, d'autant que la situation du cinéma français, je pense être en tout cas sous une grosse inquiétude après certaines déclarations, les déclarations du président de la République sur l'audiovisuel français comme un fort soutien deviennent publiques, notamment l'industrie du cinéma, donc moi je soutiens cet amendement parce que je pense qu'il y a quand même des questions qui vont se poser sur l'avenir du cinéma français de la production du cinéma français, si on remet en cause notamment le le financement et le mode de fonctionnement, le public.

Qui est contre. Abstention. Donc, l'amendement est adopté. Le 282 toujours, Madame Dumas. Merci monsieur le président, j'espère qu'on aimera plus le théâtre, encore que je remercie tous ceux qui ont adopté cet amendement précédent alors là il s'agit en effet d'un dispositif qui, de cris d'énormes pots qui est déjà en place pour différents secteurs artistiques notamment le spectacle vivant, musical, les eaux phonographique, l'audiovisuel, la création de jeux vidéo etc et cet amendement vise donc à réparer un oubli et consentir enfin au théâtre, un dispositif attractif déjà consenti à d'autres activités culturelles de création, la mission d'étude et d'évaluation, évoquée par le ministère à l'Assemblée nationale pour rejeter un amendement similaire qui a été déposé par le député de Paris, Pierre-Yves Bournazel ne peut justifier un éventuel report d'intégration du théâtre dans dans le dispositif existant, notamment parce que cela signifierait sans aucune logique que l'aide à l'émergence artistique au Théâtr serait-elle dépendant d'un bilan ministériel dans le théâtre ne serait en aucun point partie prenante l'inverse, l'intégration du théâtre à ce dispositif fiscal qui concerne principalement les nouveaux artistes en phase de développement professionnel sera une aide précieuse à la préservation d'une diversité de l'offre de création au sein du théâtre privé qui évoluent ces dernières années, vous en conviendrez tous dans un contexte particulièrement difficile, ainsi il apparaît nécessaire, dans un souci d'égalité de traitement de simulation de la création et de développement nouveaux talents d'ouvrir cette possibilité OTA privé qui je vous le rappelle représente 50 pourcent de l'activité du spectacle vivant en France. Merci l'avis de la commission, le rapporteur général. Contrairement au cinéma, d'autres parlait, c'est vrai qu'il n'y a pas de crédits d'impôt pour le théâtre et c'est un peu une exception parce que quand on regarde en effet le secteur culturel en France, il y a un très grand nombre de crédits d'impôts, ils ont été cités, cinéma, les jeux vidéo pendant des spectacles le du visuel les phonographique le spectacle vivant, les variétés, etc, etc, j'en oublie peut-être et donc, par exception dans le spectacle de la création, il semblerait qu'en effet le théâtre soit un peu l'oublié de ces dispositifs donc c'est le le raison pour laquelle on a une certaine bienveillance

merci la vie du gouvernement, on a le ministre. Si le président, monsieur le rapporteur général, je n'ai pas d'assise du théâtre annoncée, mais si vous le proposez, je peux m'engager à examiner la demande avec ma collègue de la culture très, très sérieusement,

le mécénat pour les activités de spectacles vivants et est autorisé sous la seule réserve d'une gestion désintéressée, ce qui est une une ouverture qui est favorable en effet à l'activité des théâtres et contenu du fait que le dispositif a été adopté il y a moins 2 ans, nous considérons que, l'amendement est prématurée et nous le nous en proposons le retrait. Très bien au niveau, explications de vote Madame Goulet. Monsieur le Président, Madame le Ministre, moi je vais soutenir cet amendement, contrairement à l'autre pour des raisons multiples, d'abord, il a été parfaitement exposé, le président de la a aussi justifié la sagesse, mais moi ce sera. Plutôt un vote et je vais vous dire pourquoi la fin ou la diminution des moyens des collectivités territoriales des régions, des départements qui ne peuvent plus subventionner, qui est un festival, on a vu ça déjà l'été dernier, donc je pense qu'il va falloir d'une façon ou d'une autre compenser la création artistique, également en région, parce qu'on est aussi là pour ça et et je pense que les dispositions prévues par cet amendement serait probablement un moyen de de compenser le manque de moyens dont disposent des collectivités pour aider précisément à l'offre culturelle, donc moi je soutiendrai cet amendement. Très bien, pas d'autres explications de de vote, donc je le mets au voix avec un avis de sagesse, mais plutôt favorable de la commission, une demande de retrait du gouvernement. Donc, l'amendement est maintenu, je suppose, voilà donc il est pour. Les comptes. Abstention donc l'amendement est adopté. L'amendement maintenant 722 présenté par le gouvernement. Merci monsieur le président, L'article 2 quater adopté en première lecture par l'Assemblée nationale avait élargi le Champ de la réduction d'impôt sur le revenu, accordée au titre des dons faits par les particuliers aux fondations d'entreprise en étendant son bénéfice, à compter de raconter des dons réalisés en 2017 aux mandataires sociaux sociétaires actionnaires et adhérent de l'entreprise fondatrice ou des entreprises ou des entreprises du groupe auquel l'entreprise fondatrice appartient la mise en oeuvre de de cet article de cette disposition dès 2018 aurait constitué un effet d'aubaine pour les versements réalisés en 2017 afin de l'éviter, l'article 2 quater a été supprimé en première lecture au Sénat en vue d'une adoption en seconde partie, afin que celui-ci s'applique aux revenus de l'année 2018, telle est l'objet du présent amendement. L'avis de la Commission, monsieur le rapporteur général favorable. Oui favorable de la commission, pas de d'explications de vote sur cet amendement du gouvernement qui a un avis favorable de la commission qui est pour.

Et le suivant Madame ne remédie au monsieur Baeza. Monsieur Baeza. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre Monsieur rapporteur général, mes chers collègues, il s'agit de reporter la fin du dispositif Censi-Bouvard à 2002 2018 à 2021, dans un souci de cohérence avec les dispositifs dispositions relatives aux mesures dites PTZ Pinel cette prorogation contribuera à apporter de la stabilité aux professionnels et de la confiance aux ménages investisseurs en effet la fin de ce dispositif, déjà restreint l'an passé aux seules acquisitions de logements au sein de résidence pour personnes âgées ou handicapées ou de résidence pour étudiants risque de stopper la construction de plusieurs dizaines de milliers de logements étudiants sur la mandature, allant des facto à l'encontre de l'ambition gouvernementale afin d'éviter de complexifier davantage parcourt des étudiants après la baisse des APL qui va les impacts et déjà la pénurie de logements qui résulterait de la suppression de ce dispositif risque d'accroître leurs difficultés à se loger, il convient d'anticiper la pénurie de logements étudiants qui en résulteraient, et par conséquent de déployé dispositif permettant de gérer les défis démographiques en nombre d'étudiants, ainsi, il apparaît que le dispositif Censi-Bouvard est plus avantageux pour les investisseurs les plus modestes, enfin, le dispositif dit Censi-Bouvard donne olmero meublé non professionnel, l'Avantage de déduire directement le montant de leur impôt plutôt que de leurs revenus imposables. Merci donc sur cet amendement, l'avis de la commission. L'article 39, lequel obtient s'étant déjà prolonge d'un an déjà le dispositif Censi-Bouvard qui va s'arrêter le 31 décembre 2017, il va être prolongée jusqu'au 31 décembre 2018 avec à rapport d'évaluation au 1er septembre 2018 donc, plutôt que de prolonger à nouveau pour plusieurs années, je crois que le plus sage serait datant l'évaluation au 1er septembre 2018 et je vous annonçais un scoop, il y aura une loi de finances pour 2019, il aura lieu après le 1er septembre 2018, donc nous pourrons dans le cas de cette loi de finances, examiner la pertinence de prolonger ou non le dispositif, donc je crois que vous lui attend de manière un peu donc ce ce ce, ce rapport, regardez ce qu'il en est Guy et ensuite le Sénat, le Parlement décidera s'il y a un nom de lieu de prolonger Censi-Bouvard mais avant de le faire sans évaluation, ça me paraît un petit peu prématurée, donc c'est plutôt une demande de retrait. L'avis du gouvernement. Oui, même avis pour les mêmes raisons. Très bien monsieur. Oui, ces arguments sont en effet tout à fait recevable, je m'en remets à la sagacité du rapporteur général et je donne rendez-vous donc dans un an pour le projet de loi de finances 2019.

Encore un article important de de ce PLF sur le CICE, le coût du CICE est élevé pour les finances publiques 1,7 milliards d'euros, et en même temps c'est un dispositif utile pour réorienter le comportement des ménages vers une attitude plus plus écologique donc cet article proroge le CICE en en 2018 et en le recentrant pour éviter des effets d'aubaine qui ont été bien décrit par plusieurs rapports, y compris ceux de l'ADEME, on ne peut pas suspecté d'être critique par rapport au dispositif écologique et l'ADEME montrait notamment par exemple que pour réduire d'un mégawatt, il fallait 1300 euros de cité sur les les vitres, alors que pour l'équivalent, c'était 100 euros d'isolation des toitures, donc il y a des dispositifs qui sont plus efficaces que d'autres et on sait aussi que ça a pu financer des portes blindées, par exemple, qui relève plus quand même d'une demande de sécurité ou bien des chaudières au fioul dont la performance est critiquée, donc il faut à la fois proroger le citer parce que c'est utile, et en même temps le le recentrer et c'est ce qui est fait par exemple les parois vitrées seront toujours éligible à un taux de 15 si elle remplace un simple vitrage, c'est-à-dire qu'il faut inciter à un vrai changement de comportement, on remplace un intime de vitrage par par un autre, le gouvernement s'est fixé des objectifs très ambitieux en matière écologique, notamment la réduction de 20 20 pourcent des consommations énergétiques d'ici 2030, par rapport à 2012 pourcent d'ici 2050 par rapport à 2012, donc il y a des efforts importants qui doivent être faits, mais il faut trouver les dispositifs les plus efficaces, et notamment la vraie réforme importante du CICE c'est en 2019 lorsqu'il sera transformé en prime immédiatement perceptible plutôt que un an après, parce que le frein au comportement écologique pour les ménages les plus modestes, c'est bien d'avoir avancé les travaux quand vous devez avancer les travaux ça vous dissuade alors que si vous vous dites que vous allez percevoir une prime au moment où vous les faites, hé bien vous êtes davantage incitées à les faire, donc à la fois pour corriger les effets d'aubaine et pour améliorer le comportement écologique des Français, nous avons besoin d'une réforme du CIC merci beaucoup. Merci donc sur cet article, j'ai 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Nous avons beaucoup d'amendements sur l'article 39 avec des positions parfois certains sont incompatibles entre eux, ils vont tous dans le sens de l'élargissement ou d'une prolongation, bien évidemment, je voudrais vous donner en quelques instants, la la position de la commission des finances, pas sur chaque amendement, mais au moins sur cette sur le CTE, qui vous le savez, représente un coût extrêmement important pour les finances publiques et avait il y a d'ailleurs lieu à une enquête de la Cour des comptes à la demande d'admission des fûts des finances enquête qui portait sur l'efficience des dépenses fiscales en matière de développement durable et le cette enquête a démontré que le CICE offrait un certain nombre de, avait permis, notamment, des compagnies de montée en charge des la gamme des 2 organes de la performance d'âge des équipements, mais que le CICE présentait plusieurs inconvénients, outre son coût, il était notamment peut ainsi, pour les gros travaux, il y avait des effets d'aubaine tout ça avait était signé dans le rapport de la Cour des comptes de la paix de la Cour des comptes qui avait donné lieu à une progression en commission des finances, alors dans l'attente de la transformation du CTE en prime en 2019, ce que nous repose l'article nous avons examiner, c'est le recentrage du CDE, notamment avec des dépenses qui concernait les portes, les fenêtre s'et les volets isolants qui vont être exclus du périmètre du CIT au 1er janvier 2018 ainsi que les chaudières à fioul à haute performance énergétique évidemment des combats fin dispositif il y a des mesures transitoires et c'est là-dessus qu'il y aura, il y aura, nombre d'amendements qui vont tenter d'étendre la période transitoire puisque les prêts dispositif qu'il est initialement prévu, c'est à 18 il transitoire de 6 mois entre le 1er janvier et le 30 juin et le 30 juin 2018, avec un taux réduit de 30 à 15 pourcent pour les dépenses de fenêtre et pour lui, le chat, dire au fioul et au 1er juillet 2018, à l'issue de ce dispositif transitoire ces dépenses de fenêtre s', dépenses de chaudière fioul seraient donc totalement est-ce que du bénéfice du périmètre du CTE alors je voudrais avant qu'on vote ces amendements au on se prononce sur chacun d'entre eux à rappeler quand même qu'en terme de coût pour les finances publiques, c'est une montée qui est exponentielle, puisque le coût du c'était ça presque triplé entre 2014 et 2000 16 ans 10014 c'était 619 millions d'euros le coût, et nous en sommes maintenant à un milliard 7 puisque, notamment, il y a eu un taux unique de 30 pourcent donc ils font attention à l'expansion de ces dépenses fiscales dont l'efficacité est parfois sujette à caution et jour si vous en voulant savoir plus regarder à nouveau l'enquête de la Cour des comptes à la et commissions des Finances

pourcent d'objectifs sur la période 2009 2016 aucune efficacité limitée, un coût pour les finances publiques important donc, soyons très prudents face aux demandes d'extension de prolongation et heureusement pour laquelle la commission des Finances jeudi par anticipation par rapport aux différents un moment pour l'écarter de débat va être assez réservée ou défavorable aux amendements d'extension avec une sagesse plutôt bienveillante sur le 271 272 et sans doute de 73, donc ils sont des 18 if très limitée et très ciblée sur la transition, mais ce sera sans doute beaucoup plus réservés sur les autres dispositions.

Alors certes, Monsieur le, le rapporteur général, vous, vous le disiez le le CIT représente un coût important pour les finances publiques cependant sur bon nombre d'indicateurs, nous sommes en retrait en deçà des objectifs que nous avons pourtant validé de manière très importante, très éclatante au moment de la de donc certes il convient peut-être de de repositionner un certain nombre de, de, de dispositifs sur des choses qui sont vraiment efficaces en terme énergétique mais cela dit,

une vision globale de la situation de leur logement pour permettent de faire le bon diagnostic et donc les bons travaux et je pense que c'est ce ce, ce sur quoi il faut s'orienter, afin que le CICE soit vraiment efficace, en terme énergétique et que nous puissions relever le défi de la transition énergétique du chômage. Pas d'autres prises de parole sur l'article 2 donc sur l'amendement 211 Madame de remédie. Oui, merci Monsieur le Président, contenu des explications, monsieur le rapporteur, je vais retirer cet amendement au profit des amendements 271 et 272. Alors donc c'est noté donc dans la discussion commune j'avais également un amendement. Monsieur Beauquier. Oui, merci Monsieur le Président, d'obscénités que le gouvernement entend transformer en prime à l'horizon 2019 le concept pourrait donc changer mais les caresser les caractéristiques pardon en demeure cette démarche évidemment que nous approuvons mérite, nous semble-t-il, un effort particulier, non seulement sur le plan fiscal, mais aussi sur le plan économique le message est relativement entendu avec depuis plusieurs années aux alentours de 1000 700 millions d'euros de crédits d'impôt partagé entre plus d'un 1000000 de contribuables, il faut continuer de favoriser la réalisation de travaux d'amélioration des performances énergétiques dans les logements individuels comme collectifs d'ailleurs en tenant compte des spécificités de certains territoires et en mettant en place des financements dédiés peu onéreux pour les emprunteurs et susceptible de favoriser la réalisation d'un diagnostic complet des logements et une intervention globale, la formule de l'éco-prêt à taux 0 et son crédit d'impôt associés dans le code général des impôts semble aujourd'hui beaucoup trop confidentielle au regard du nombre de redevables qui l'ont sollicité, rappelant la portée de l'article L 221 du Code monétaire et financier qui dispose que je cite les ressources collectées par les établissements distribuant le Livret A ou le Livret de développement durable et non centralisée en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leurs créations et leur développement, ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens, ils sont forts et donc de procéder à quelques ajustements de cet article pour mettre en évidence la mise en grève de la transition écologique, une telle démarche, il faut souligner permettrait de compléter utilement un dispositif de crédit d'impôt dont le défaut essentiel et d'exiger du contribuable, une avance de frais, merci. Sur cet amendement, l'avis de la commission. Donc j'déjà évoqué à l'instant défavorable. La vie du gouvernement.

et de le rendre plus efficace. Comme vous le savez, initialement, l'article 8 du PLF proposé de tirer immédiatement soit dès l'annonce en conseil des ministres le 27 septembre 2017, les conséquences du rapport rendu par la mission IGF GED dès cette date du 27 septembre a suscité quelques incompréhensions de la part des professionnels et de vos collègues députés néanmoins après concertation, il me semble que nous sommes parvenus à un accord équilibré, qui tient compte à la fois des préoccupations des professionnels et des exigences d'amélioration de l'efficience du CTE et c'est pour. Quoi, je suis défavorable aux amendements d'extension des dates de la transition. Merci donc, si je n'ai pas d'explication de vote je mais on voit avec que 2 avis défavorables de la Commission et du gouvernement qui est pour. C'est con. Abstention donc l'amendement est rejeté. Alors nous avons ensuite. nous avons ensuite une série d'amendements en discussion commune 16 exactement. Donc, je commence par le 675.

cet amendement a pour but, tout simplement, de se mettre en phase par rapport à la réalité de ce qu'on a aujourd'hui sur le parc des chaudières fioul sur un parc de 3000 3 millions de chaudière, on a un 1000000, plus de 25 ans, avec des rendements qui sont aux alentours de 60

pour notamment les ménages les plus faibles de pouvoir continuer d'améliorer la performance énergétique mais ce qui est surtout un temps important à travers cet amendement, c'est qu'il cible les chaudières à eau à haute performance énergétique et non à très haute performance énergétique et haute performance énergétique sont aux alentours de 90 pourcent les très hautes, à 92 pourcent la conséquence si on telle que c'est aujourd'hui dans le texte on exclurait en fait l'ensemble des bénéficiaires puisque aujourd'hui l'ensemble du parc 91 pourcent des chaudières fioul françaises sont à haute performance, soit 90 pourcent de de de rendement et puis en plus ce qui est surtout le plus important, c'est le niveau de de prix 2400 euros de plus pour une chaudière entre la haute et la très haute performance, donc ce qui vous est propre proposé tout simplement c'est de permettent effectivement d'améliorer le parc des chaudières à fioul et surtout de permettre aux ménages les plus modestes de pouvoir améliorer à la fois la performance énergétique de diminuer la consommation de fioul dans notre pays, de répondre à la problématique des gaz à effet de serre et et surtout, là encore monsieur rapporteur général, j'ai bien entendu votre message puisque la proposition à travers cet amendement traduit une diminution de moitié au niveau des crédits puisqu'on passerait de 20 millions d'euros en termes de consommation à 10 millions sur les conséquences de l'application de tels amendements. Merci le 366 présenté par monsieur de la neige. Merci Monsieur le Président, cet amendement est dans la lignée de celui qui vient d'être présenté par Monsieur Gremillet qui soulève tous les problèmes d'évolution de la législation et de dates et, par conséquent, je vais me rallier bien volontiers à l'amendement qui l'a présenté au nom de la commission des affaires économiques et si on plus ça peut conforter, monsieur le rapporteur général dans la bienveillance qui l'a exprimé tout à l'heure, je ne doute pas que l'objectif poursuivi sera atteint, je vous remercie, je retire donc cet amendement. Donc je considère que le 366 et retiré. Ensuite j'ai 6 amendements identiques,

il est précisé, mais ça a déjà été dit que ce sont véritablement les ménages les plus modestes ou les plus isolés géographiquement, qui ont besoin de ce type de chaudières au fioul. Très bien, le 661 Monsieur

Madame Cosse. transition énergétique, Nicolas Hulot et le ministre de la cohésion des territoires Jacques Mézard ont présenté le 24 novembre dernier un peu ambitionne Renaud-Bray une rénovation énergétique des bâtiments, ce plan constitue une feuille de route, essentielle pour faire de la rénovation énergétique une priorité nationale, la France compte aujourd'hui 7 à 8 millions de logements considérés comme de véritables passoires énergétiques soit logement sur IV, les travaux d'isolation thermique, peuvent contribuer à une croissance économique vertueuse créatrice d'emplois dans le cadre du plan qui afin de rénover en disant un 1000000 et demi de passoires thermiques habité par des ménages propriétaires à faible revenu, le gouvernement souhaite accompagner financièrement 150000 rénovations par an cet amendement s'inscrit complètement dans cette logique en prorogeant le crédit d'impôt, transition énergétique à 15 pourcent pour le remplacement des fenêtre simple vitrage et pour les Chaudel chaudière à fioul fioul performances jusqu'au 31 décembre 2018, en effet on ne comprendraient très mal que les fenêtre et les chaudières haute performance soit exclu dès le 30 juin 2018, comme l'a proposé le gouvernement dans son amendement, adopté à l'Assemblée nationale, d'autant que le CIT eux viennent en première position des aides sollicitées par les ménages le CICE dispositif bien identifié par les ménages, en 2015, il a représenté près de 6 milliards et demi d'euros de travaux et 73000 emplois en particulier les travaux sur les fenêtre concerne le tiers des logements, le remplacement des simple vitrage représente, selon les experts, quelque 60 pourcent de ses travaux sur les fenêtre éligible au CIT concernant le chauffage au fioul, l'exclusion des chaudières haute performance risque de dissuader les remplacements de chaudière, alors que, selon l'INSEE 84,6 millions de foyers utilisent ces foyers sont souvent contraints à ce mode de chauffage en raison de l'isolement géographique du logement et surtout parce qu'il reste le meilleur marché sur les autres sources d'énergie, la proposition de cette admin on demande un coup par ailleurs raisonnable et donc cohérente avec telle que le gouvernement souhaite apporter aux ménages confrontés à la précarité énergétique et avec les objectifs de la transition écologique. Merci donc le l'amendement suivant toujours. Dans la même série Monsieur Rémy et au nom de la commission des affaires économiques. Oui, merci Monsieur le Président, on administre, monsieur le rapporteur Gérard, chers collègues, effectivement, au nom de la commission des affaires économiques, cet amendement concerne de prolonger jusqu'au 31 décembre un taux réduit de crédits d'impôts à 15 pourcent au lieu de 30 pour les fenêtre nous avons bien entendu effectivement nous excluons les les portes et volets comme ça a été notamment évoqué par notre rapporteur général mais surtout cet amendement donne un signe, un signe de performance énergétique puisqu'on diminue de 15 pourcent certes le les conséquences sur les économies d'énergie sont plus faibles qu'avec des travaux très lourd sur les toitures en particulier, mais bien plus accessible à de nombreuses familles et aujourd'hui dans la proposition, à travers cet amendement, ça permet de continuer d'améliorer la performance énergétique du bâti, ça permet de continuer : donner un signe aux familles avec des revenus modestes et ça permet aussi d'atteindre l'objectif de d'économie puisque, comme l'a souligné tout à l'heure, tout à l'heure notre rapporteur général dans cette proposition et l'application en termes de de conséquences financières, on passerait de 630 millions de d'euros avec ça permettrait une économie de 425 millions puisque on serait aux gens autour de 200 millions en terme de conséquences budgétaires donc efficacité moindre coût et surtout accessibilité aux ménages les plus faibles. Merci, alors le 400 89 qui est ce qui le défend monsieur Baeza.

donc si ces 2 amendements sont votés, celui-ci devra-t-être votée par contre si ils ne sont pas voter, celui-ci n'a pas, n'a plus de raison d'être en terme.

vous savez 2 coqs au 1er janvier 2019 il y a le système de la prime, donc ça évidemment se pose toujours la question de la période transitoire pour les raisons à la fois de coups de mesure de l'efficacité pour les raisons qui ont certaines étaient et partagez avec la Cour des comptes, à l'occasion de son rapport et du travail qui a fait la commission des finances

et par coordination le 273 donc de 71 de 72 de 73 2 collègues Gremillet, pourquoi, parce que ces 2 amendements proposent une prolongation de 30 juin au 31 décembre 2018, à la fois pour les chaudières au fioul et pour les doubles vitrages, plutôt que de s'arrêter à mi-chemin en cours d'année ça permet l'adaptation des différents acteurs au dispositif le coup on est limité et donc ne pas être raisonnables datant de 2 de pouvoir aller jusqu'à la fin de l'année pour que, encore

Madame la ministre, le l'avis du gouvernement. Comme indiqué, donc le gouvernement est défavorable à ces amendements, y compris ceux qui sont soutenus par la commission des finances. finances. Donc, je vais mettre aux voix les différents amendements s'il y a pas d'explication de de bottes Bartosz je regardais à droite et à gauche, mais pas au milieu Monsieur Delcros. Com. Mais que ces ces dispositions fiscales, ce crédit d'impôt, a bien un double objectif : un double objet : d'une part sur de de point de vue général, bien entendu, l'idée c'est de de lutter contre réchauffement climatique de diminuer les gaz à effet de serre etc, évidemment, c'est un objectif qu'on partage mais n'oublions pas que, individuellement, il permet aussi de réduire la facture des charges, le coude, chauffage, je pense notamment aux habitations qui sont situées en altitude en montagne pour des ménages à revenus modestes, et donc je pense qu'il faut dans l'eau, décision et dans nos vote avoir toujours présent à l'esprit ces 2 objectifs qui se rejoignent, bien entendu, mais qui peuvent nous allons nous amener à moment à à faire des bottes, un peu différent si on prend en compte ce 2ème objectif, qui est extrêmement extrêmement important et je veux rappeler que pour des personnes à revenus modestes, le coude chauffage en montagne est un élément extrêmement important, c'est une charge importante pour ces ménages. J'ai vraiment. Oui, Monsieur le Président, sans trop prolonger le débat, je voudrais dire tout simplement j'ai remercier notre rapporteur général de de cette position de sagesse, bon allez, je suis un peu surpris parce que la proposition, les 2 amendements. Ne crée pas de rupture. ça permet effectivement de passer du système du site à la prime 2019, et en plus les conséquences financières sont dans l'objectif puisque notre proposition va au-delà, en terme de d'économies sur 6 mois, on fait plus d'économie en enclos qu'en 6 mois, et puis la dernière remarque, on ne peut pas comme ça, laisser de côté, autant de familles avec des revenus très faibles sur la précarité énergétique et là ça contribue aussi au gaz à effet de serre. Merci, je n'ai pas d'autres explications de vote monsieur Baeza. Merci Monsieur le Président, j'ai bien sûr voter les amendements qui ont été l'objet d'un avis favorable de la commission des finances je voulais ajouter au aux 2 points qui ont été évoqués par notre collègue, un 3ème qui l'impact sur l'activité économique, parce que quand vous avez un dispositif qui s'arrêtent un trou de 6 mois et un autre qui va prendre le relais après vous allez avoir nécessairement un impact sur l'activité des entreprises qui vont avoir un trou d'air et ensuite à un trop gros pas afflux de commandes, donc ça doit être aussi pris en compte, je crois que c'est un 3ème élément ajouté. Merci donc je peux mettre aux voix le 271 avec. Un avis de sagesse favorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement sur le 271 qui est pour. Qui est contre. Abstention donc il est adopté. Et, en conséquence de 466 E 617 que 661 et le 563. Donc j'en arrive au vote sur le 272 présenté par Monsieur Rémy, au nom de la commission des affaires économiques. Est ce qu'il a des explications de vote, pas d'explication de vote donc avec un un avis de sagesse. Favorable de la commission est défavorable du gouvernement le 272 qui est pour.

ça, la maman de coordination. Alors ensuite 2 amendements identiques en discussion commune. Le 1er n'est pas soutenu et le second Madame polluant. Merci Monsieur le Président, Madame la ministre, cela a été dit, les enjeux climatiques majeurs auxquels nous faisons face et les engagements pris à l'occasion de la COP 21 nous impose d'agir pour sortir la France des énergies carbonées et de développer un large éventail de solutions renouvelables alors c'est vrai, les portes blindées ne répond pas à ces objets. Chiffre mais la chaleur solaire fait partie de ces solutions en offrant à vecteur performant de chaleur renouvelable pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire place de ce constat, pardon la programmation pluriannuelle de l'énergie affiche des objectifs ambitieux en la matière, bien qu'elle bénéficie d'un soutien au travers du crédit d'impôt du crédit d'impôt, transition énergétique, les installations chauffe-eau solaires sont en berne, bien en deçà de la trajectoire inscrite au PPE, les estimations que nous avons aujourd'hui montrent que seuls 10 pourcent de l'objectif pourrait être atteint en l'état actuel des choses, donc cet amendement propose de permettre que la pose de ces équipements puisse également entrer dans le périmètre du crédit d'impôt, comme cela se fait pour l'isolation ou le forage depuis géothermique en effet la part de main-d'oeuvre représente aujourd'hui 25 à 30 pourcent de la fin. Sur finale du consommateur et demeure un frein majeur pour nos concitoyens, donc l'inclusion de la pause dans le périmètre du CICE permettrait d'offrir un signal fort et de soutenir l'artisanat local, en effet, ces technologies demande une main-d'oeuvre qualifiée local bien sûr et non délocalisables cette inclusion de la Main-d'oeuvre resterait bien évidemment encadré par le plafond réglementaire qui s'applique à ces technologies pour éviter les effets d'aubaine sans un véritable coup d'accélérateur, un véritable portage politique un signal clair envoyé aux consommateurs la PPE restera lettre morte, déclaration de bonnes intentions, bien loin du document stratégique, elle est censée être et, donc, cet amendement vise à y remédier je vous remercie. Merci l'avis de la commission. C'est un petit peu contradictoire avec l'objectif de resserrer le crédit d'impôt la puisqu'on irait vers une exception serait plus le coût de l'équipement, mais également à la manoeuvre, là au outre le fait que c'est une exception au principe général qui veut que les frais annexes soient pas pris en charge, je pense que ça pourrait poser des problèmes techniques ou d'appréciation puisque quand vous et le coût d'équipements, vous avez la facture, vous savez combien coûte une c'est-à-dire un chauffe-eau si on se met avec la devra quelqu'un refait une salle demain, quelle est la part afférentes au seul coût de pause du chauffe-eau, donc ça peut donner lieu à toutes sortes de d'abus d'interprétation donc son avis défavorable. L'avis du gouvernement. Oui, merci Monsieur le Président, lorsque, comme ça été rappelé la règle générale et d'exclure les dépenses de main-d'oeuvre pour concentrer le soutien public sur les équipements le gouvernement est défavorable à cet amendement. S'agissant de la pose des équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable et au cas particulier des pompes à chaleur géothermique, le dispositif est déjà favorable puisque les travaux de pose de l'échangeur de chaleur souterrain de ces dernières ouvrent droit depuis 2010 au crédit d'impôt du Fedor poids dans la dépense, dépense globale, il n'y a pas lieu d'état d'étendre cette dérogation aux dépenses de la pompe à chaleur elle-même.

on a fini un CAP de transition énergétique et comme par hasard, on découvre, on n'atteint pas. Et on trouve toujours, mais alors là, ça fait des années, des années 25000 arguties techniques pour nous expliquer qu'il faut pas, il y aurait de la dérogation, il y aurait des trucs, c'est tellement compliqué. C'est tellement restrictif que premièrement une large partie des gens peuvent pas faire les travaux, deuxièmement, qu'on sait jamais sur quel crédit d'impôt, on peut, on peut compter où, sur quelles aides on peut réellement compter et bilan des courses : la France est en retard par rapport à ses objectifs, on est tous en train dire qu'on a un problème d'emploi. Et qu'est-ce qu'on enlève dans les dépenses. Les frais de main-d'oeuvre dont je vous rappelle que les maîtres c'est aussi invité du travail au noir, les maîtres c'est aussi pousser les artisans à former davantage une main-d'oeuvre nationale et pas faire appel au coup par coup à une main-d'oeuvre venant d'un en travailleurs détachés, donc franchement à la fois du point de vue de la structuration de la filière, à la fois du point de vue de l'efficacité au regard de nos engagements, comme 21 et comme l'ont très bien dit, certains collègues au regard de la de la amélioration du pouvoir d'achat, ça constitue avec un allégement des charges et enfin de l'emploi, je trouve que là, on fait des économies de bouts d'chandelle ou quand on fera le bilan global et ben la nation c'est retrouverait donc moi je j'appelle les collègues à voté pour cet amendement. D'autre explications de vote, donc je vais mettre c'est amendements aux voix avec 2 avis défavorables. Qui pour.

Oui, Monsieur le Président, cet amendement vise à étendre le CIT aux pompes à chaleur géothermique elle-même aujourd'hui l'échangeur souterrain est éligible, mais pas la pompe elle-même, comme il s'agit d'un équipement et non pas de la pause, ça répond à la demande de la ministre, qui indique que ce sont les équipements qui sont soutenus, donc je vous propose, compte tenu du marché important et du coût que ça représente pour les foyers d'introduire la pompe à chaleur géothermique elles-mêmes dans l'éligibilité. aujourd'hui, l'article 10 de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermique, je vous propose de remplacer par les mots des pompes à chaleur géothermique et leur échangeurs souterrains.

des pompes à chaleur et j'ai entendu ce qu'a dit Madame Neeman la Madoff n'a jamais été prise en compte donc c'est pas une restriction de ce point de vue, on a toujours pris en compte le coût des équipements jamais la Main-d'oeuvre ça coûte déjà un milliard 7 et si on prend la main d'oeuvre, je pense que ça peut poser préoccupent, problèmes de périmètres parce que autant le coût d'équipement, vous avez une facture, vous savez qu'une pompe à chaleur à chauffe-eau coûte tant ou tant sur la Main-d'oeuvre lorsqu'on voit les travaux divers et variés, la tentation sera évidemment d'affecter plus de Main-d'oeuvre sur la pose des équipements qui sont les peu d'impôts, donc, pour les raisons que j'expliquais ces ces défavorable et s'introduire en tous les cas une exception au principe général que les frais annexes, notamment la Madame ne sont pas pris en compte. Il y a là l'avis du gouvernement, le ministre. Défavorable également. Donc pas de

Qui est contre. Donc ils ne sont pas adoptées. 2 amendements identiques, le 515 n'est pas soutenu. Le 662 Madame polluant. Monsieur le président, Jean merci alors là, je vais peut-être avoir davantage de succès puisque, effectivement, personne ne s'oppose au fait qu'il fallait bien centré ses aides sur des choses qui sont je dirais vraiment efficace, je dirais, participer à un certain nombre d'abus et c'est ce qu'on observe en particulier en ce qui concerne les chauffe-eau thermodynamique cette technologie permettant de produire de l'eau chaude à partir des calories présentes dans l'air environnant, offre une solution économique, écologique, intéressantes, mais on constate que s'échauffe au terme thermodynamique sont vendus isolé ment à des prix très élevés ou associé à d'autres produits non éligible pour atteindre le plafond du crédit d'impôt, tandis que le prix catalogue de ses équipements et située entre 2 et 4000 euros, dès lors, poursuivant un objectif de bonne gestion des deniers publics qui est largement partagée sur ces cet cet amendement vise à plafonner le CIT pour les chauffe-eau thermodynamique afin de mettre fin aux abus et aux effets d'aubaine constatés comme cela existe pour les équipements, chauffage et d'eau chaude solaire depuis 2009 une modération des dépenses consacrées à ces chauffe-eau permettrait de limiter de 20 à 50 millions d'euros, les dépenses de CTE et cela permettra permettrait aurait permis de prendre en compte un certain nombre d'autres dépenses qui elle serait mieux ciblées, je vous remercie. Oui, donc l'avis de la commission. Je jusqu'un peu puisque lorsqu'il y a un Avantage fiscal, ça peut être inflationniste et à conduire le consommateur à à surpayer un équipement dans la mesure où évidemment les vendeurs de ces équipements ne sont pas idiots ont bien compris qu'il vendait à prix avec l'Avantage fiscal et dans ce package, ils ont tendance à augmenter leurs marges et le prix de l'équipement, alors peut-être qu'il y a des abus sur telle ou telle petite d'équipements donc l'idée que l'on a un peu référentiel fixé par voie réglementaire, est une idée plutôt saine et donc le le le climat favorable ces monuments. Oui, Madame la Ministre. merci monsieur le président, le le objectif de plafonnement vertueux bien évidemment, donc nous y souscrivons on a eu un petit débat parce que il nous semblait que la mesure était un peu vaste, et pas forcément simple à appliquer, il faut, il faut des systèmes de plafonnement qui soit suscite suffisamment précis précis pour ne pas être des incitatifs ou ne pas créer justement de les effets qui aille à l'encontre de l'objectif, voilà, ça n'a pas été expertisée au bénéfice de la, de l'objectif vertueux de la mesure, je veux dire sagesse.

le gouvernement s'était à l'époque, engagé, n'ont pas créer un observatoire parce que c'est très lourd, mais avec, notamment, dans la commission où sont tous les ans, les professionnels du secteur et, notamment, du bâtiment et des économies d'énergie, il avait été prévu de faire une analyse de l'évolution des coûts des différents produits des différentes méthodes de d'isolation ou d'énergies renouvelables et de comparer cette évolution des cours aussi avec les évolutions des coûts dans les autres pays de l'Union européenne pour qu'on ait pas s'était fait que monsieur De Gaulle Montgolfier vient de d'indiquer, à savoir des dérapages et des augmentations qui absorbe les crédits d'impôt. Je voudrais demander au gouvernement s'il avait l'intention de continuer un travail d'ou de mettre en oeuvre un travail de cette nature, Merci donc pas d'autres, les explications de vote, donc je peux mettre, je peux mettre aux voix avec un avis favorable de la commission et sagesse du gouvernement qui est pour.

Pour le 637. visant à étendre le Champ d'application du CIT aux prestations de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux proposés dans le cadre de l'eau dite énergétique qui garantira leur mise en oeuvre et un suivi par des professionnels compétents et assuré à ce titre-donc comme je trouve cette avec monsieur Sueur nous avons trouvé cette demande légitime cette proposition intéressante, nous leur soumettons. Merci donc le le suivant identique le 709 qui a défendu par. Alors j'ai le choix monsieur Baeza monsieur et qui s'est absenté madame de remédier. Défendu si identique donc le 709 et défendu avis de la Commission sur ces 2 amendements identiques.

aller jusqu'au prestation de maîtrise d'oeuvre, ça semble surabondant et donc c'est un jour de l'avis défavorable. Madame la Ministre. Mais magique. Avis défavorable, donc je peux mettre aux voix, pas d'explications de vote. Donc avec enfin. Papa réservé quasiment défavorable ou très réservée de la Commission un défavorable du gouvernement qui est pour.

Oui, je vais essayer d'être un peu plus clair que tout à l'heure parce que effectivement dans l'amendement précédent le rapporteur général Aral avait raison, je parlais bien de la poser cette fois-ci je vous parle de la visite préalable à l'installation ou à la pose des équipements ou des matériaux objet de cet amendement propose de permettre à l'entreprise recourant à un sous-traitant pour l'installation ou la pose des équipements qu'elle fournit d'effectuer elle-même la visite préalable à l'installation en effet aujourd'hui en raison de la forte saisonnalité des ventes de nombreux fabricants français sont obligés de sous-traiter la pose de leur équipement à des artisans locaux cette proposition répond donc à une réalité du marché et vise à mettre fin à un blocage technique. Alors les 2 autres amendements, discussions communes sont qui ne sont pas défendus, donc je vais demander l'avis de la commission.

Avis du gouvernement. Oui, de demandes de retrait également. Je pense que la la qualité de l'installation est assurée par l'entreprise qui installe et qui pose, il est donc légitime que ce soit l'entreprise qui va exécuter les travaux et je, je, je rappelle qu'il y a une cohérence du dispositif avec une

Merci donc demande de retrait monsieur qui a plus de demandes de retrait, vous maintenez. Maintenu donc je mets au voire avec 2 demandes de retrait de la Commission et du gouvernement. Mais pour. Qui est contre. Abstention donc il n'est pas adopté, je mets ou voit maintenant l'article 39 Denise. Qui est pour.

pour qui ces questions sont particulièrement importantes, donc c'est effectivement la vente de chaleur, faire en sorte qu'elle puisse l'énergie solaire thermique étant par essence une source renouvelable de chaleur, il convient donc de la pure explicitement dans le calcul de la part d'énergies renouvelables, ouvrant droit au bénéfice du taux de 5,5 Très bien, donc, sur ces amendements la de la commission.

Alors. Certes, l'extension du taux réduit de la TVA la fourniture de chaleur produite à partir d'autres sources d'énergie renouvelables et souhaitable dans une logique incitative environnementale, toutefois, telle que proposée l'amendement aurait pour effet d'organiser une cannibalisation de certaines sources d'énergie par d'autres, en effet, l'extension du dispositif à une nouvelle forme d'énergie pourrait conduire au remplacement des énergies renouvelables renouvelables déjà prise en compte par le dispositif en vigueur, il conviendrait donc avant d'envisager une extension du taux réduit de la TVA de réexaminer la pertinence de l'ensemble du dispositif, notamment s'agissant de la proportion minimale d'énergie renouvelable, à partir de laquelle les réseaux sont éligibles, je vous propose donc que le gouvernement conduit les travaux en ce sens et que vous nous y revenions ultérieurement, et donc je vous propose le retrait. Bien donc demande de retrait du gouvernement est-ce que les amendements sont maintenues, monsieur rénale. Nous sommes dans la discussion législative, ça s'appelle madame la Ministre, la navette, donc moi je propose qu'on le vote et que vous réfléchissiez que vous Très bien, donc monsieur qui est plus non plus, donc les amendements sont maintenues, j'ai. Pas d'explication de vote. Qui est pour.

Alors, cet amendement, je crois qu'il est unique, il vise à clarifier le régime fiscal applicable aux installations d'énergies marines renouvelables EMR en alignant leur régime sur le régime assuranciel des véhicules maritime, il prévoit notamment d'étendre l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance dont bénéficient déjà les véhicules maritime aux installations d'énergies marines renouvelables, la mise en place d'une telle exonération contribuerait à faire baisser les coûts de la filière des OMR et accompagner le développement de nouvelles formes d'énergies renouvelables en France, cet amendement mais en cohérence la fiscalité relatives aux conventions d'assurance avec l'évolution introduite par la loi du 20 juin 2016 pour l'économie bleue. Si David la Commission, monsieur de Montgolfier. à priori, c'est une perte de recettes de la taxe sur les conventions d'assurance, c'est un produit pour les départements, alors en mer, il faudrait vérifier avec préavis du gouvernement, par définition n'est défavorable à cette perte de recettes et de gouvernement ne peut nous expliquer sa position sur cet amendement, qui avait rejeté à l'Assemblée nationale, avec une absence d'explication qu'il n'y a pas beaucoup éclairé le Parlement. L'avis du gouvernement, Madame le Ministre.

merci Monsieur le Président, donc la loi pour l'économie bleue du 20 juin 2016 à rapprocher le régime assuranciel des installations d'énergies marines renouvelables de celui applicable applicable aux coques de navire, les installations d'énergies marines renouvelables relève depuis la depuis de la catégorie des grands risques au sens du code des assurances et donc le gouvernement est favorable à cet amendement qui en tire toutes les conséquences en matière de taxe spéciale sur les conventions d'assurance. Oui, madame la ministre, si vous êtes favorable, vous êtes favorable d'accord pour lever le gage. Oui, oui, d'accord. Très bien sur cet amendement 255 est ce qu'il y a des explications de vote. Non, donc je vais le mettre.

D'accord, demande d'avis du gouvernement, donc la Commission suit l'avis du gouvernement, donc avis favorable du gouvernement et de la Commission. J'ai mis aux voix qui est pour. qui est pour. Comptes. Abstention donc l'amendement est adopté. Alors les amendements en discussion commune 5 amendements. Le 1er n'est pas défendu 496. Ensuite le 584 Madame Goulet. Monsieur Président, même le ministre cet amendement à un objectif extrêmement précis et en plus c'est un problème extrêmement concret, il s'est d'ailleurs produit dans mon département une perspective d'implantation. Andéol yen dans un territoire, il est prévu un mécanisme incitatif sous forme d'une attribution de 20 pourcent de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau cette par constituer également une compensation des éventuels le désagrément causé par un parc éolien et puis aussi des travaux et des marques qui ont pu être accomplis par les différentes collectivités, de façon à à traire ses ces éoliennes sur leur territoire, or les communes qui accueillent des éoliennes ce ne se voit pas reverser une part des recettes de l'faire, en effet, dans le cas où le PC d'appartenance à opter pour une fiscalité professionnelle unique, ce dernier perçoit la totalité du produit du produit l'hiver éolien sans aucune obligation de reverser une partie à la commune d'implantation et si vous ajoutez les modifications de la loi nôtre si vous me dites si vous ajoutez tous les toutes les modifications des périmètres, vous voyez qu'un certain nombre de communes qui, dans le cas d'une intercommunalité ou ont installé des éoliennes se retrouvent absorbé dans une autre intercommunalités qui va bénéficier de l'ensemble des revenus de ses éoliennes sans leur reverser une partie alors que ce serait tout à fait normal puisque c'est elle qui ont fait d'investissements à la fois en temps et en énergie, et c'est le cas de le dire, donc, les communes sont donc de moins en moins incités à accepter des projets éoliens, cet amendement vise donc à ce que toutes les communes d'implantation puissent bénéficier de l'hiver, éolien, quel que soit le type de PCI d'appartenance. Merci, on continue la discussion commune avec le 256 monsieur a pu. Oui, il est défendu, c'est la même logique que celui qui vient d'être défendu par Madame Goulet.

Alors, lorsque les faire a été créé il y a eu de très longs débats ici, je me souviens, sur la répartition du produit, de les faire entre les communes, les EPCI, les départements, c'était des soirées extrêmement pénible, longue autoroute ça brasser beaucoup d'air assez normal pour des éoliennes et en tous les cas, on est parvenu à l'issue de ces longs débats, ce qui ne semble une position d'équilibre si on adaptait ces amendements ça modifierait l'équilibre dans les ressources à un moment où il y avoir des débats importants jeudi prochain et la conférence des territoires et il y aura des dispositions dans la loi de programmation des finances publiques sur les ressources des collectivités et donc est-ce que c'est le moment très concrètement d'aller modifier l'équilibre qui a été atteint, notamment sur la peau, le rire parce on l'y faire, c'est pas la position de la commission d'autre part, si on a peu de pièces amendement, il y aurait eu une incohérence, par exemple, je prends l'exemple d'une centrale nucléaire,

donc il y aura un problème de logique de répartition de lier, de les faire avec d'autres formes d'énergie, ça crée un régime spécifique sur la vie, ce qui a été éoliennes qui serait différent de celui des autres installations en matière d'énergie, donc c'est une demande de de de retrait ou un avis défavorable sur ces amendements. Oui, Madame la ministre du gouvernement. Oui, merci Monsieur le Président, de notre côté, c'est également une demande de retrait. Car cette proposition va à l'encontre de l'intercommunalité et déroge au principe de la fiscalité unique n'incite pas les collectivités assiégée vers plus d'intégration fiscale alors que l'objectif sous-jacent, et de les inciter à agir au profit de l'intérêt communautaire. Au surplus, les OPC en question verse déjà aux communes concernées, une fraction de leurs ressources due à une attribution visant à compenser les nuisances liées aux installations éoliennes donc demande de retrait sinon merci. Merci

questions des collectivités territoriales, je, je, je suis pas sûr qu'il faille touchés par le PLF ces questions-là, je pense qu'on fait toujours plus de dégâts qu'autre chose, en essayant de modifier à travers le PLF des

et si ça va pas aux communes, hé bien les communes s'arrêteront alors si on tient ce raisonnement, ça vaut pour tout le tout le domaine économique, lorsque vous avez aujourd'hui une entreprise qui s'installe, la commune, elle reçoit certains la taxe foncière, mais tout le reste va à l'interco et c'est pas un sujet, ce n'est plus le sujet donc je vois pas bien pourquoi il y aurait une spécificité effectivement au niveau de l'éolien, je trouve que c'est pas très bon, et moi j'encourage aurait plutôt les interco être effectivement le plus intégrée possible et ensuite à faire jouer éventuellement si elles le souhaitent, des dotations de solidarité communautaire qui peuvent tout à fait naître, qui est un angle, un des éléments, soit par exemple le fait d'accepter des éoliennes sa commune, ça peut être tout à fait un élément d'une dotation de solidarité communautaire bien conçu, donc moi j'invite à l'Intelligence collective au niveau des territoires et je voterai pas cet amendement ces amendements. Madame rouler. qui est le 1er signataire et qui considère aussi que l'incitation fiscale dans ces cas-là, peut-être important pour ces énergies renouvelables, mais moi je, je voudrais préciser qu'effectivement, quand vous avez une je je parle en terme de de révision notamment sud à la suite de la loi nôtre, c'est-à-dire de l'intégration d'une intercommunalité tu dois tout allait très bien, rentre dans une autre intercommunalité et ce petit noyau de l'intercommunalité absorber ne perçoit plus aucun ben j'entends, j'entends bien ce que vous dites donc vous dites une une péréquation intelligente à l'intérieur de la ville de l'intercommunalité, mais si elle n'existe pas ou si elle ne se fait pas

je vais donc retirer cet cet amendement mais je voudrais, je voudrais quand même dire que dans dans un cadre ou dans un autre, il faudra probablement revoir comment on travaille sur la péréquation à l'intérieur des nouvelles intercommunalités reconstitué à la dans le cas de la loi, note parce que vous avez quand même des communes qui ont fait énormément d'investissements qui sont absorbées sans plus jamais recevoir le bénéfice du travail initial qu'elles ont fait, donc c'est sûrement par le biais de la péréquation et de l'Intelligence territoriale dans le territoire ne manquent pas et donc je vais retirer cet amendement.

veux je veux juste apporter un autre élément d'un dans dans la réflexion sur cette question des éoliennes, c'est que là on vise finalement à permettre à la commune sur laquelle sont implantées les éoliennes de bénéficier davantage de retombées par par l'hiver, mais l'impact des éoliennes ne concerne pas seulement la commune sur laquelle sont implantés et même parfois l'impact est plus important pour des communes limitrophes que pour la commune pour la sur laquelle elle sans centaines plantées, donc je trouve que l'approche intercommunal et pour à la fois pour régler pour régler la question des retombées fiscales mais aussi pour régler la question des compensations éventuelles en fonction de l'impact, qui peut être donnée, notamment en terme de de paysage nuisances à l'implantation des éoliennes.

par la réflexion qui est nécessaire parce que les Chamois éoliens qui sont mis en place depuis quand même maintenant pas mal d'années il faut du temps aussi pour implanter des éoliennes et on voit la complexité dans le cas des déchets Véolia en prêt il y a les les retombées financières naturellement que alors il y a des communes et c'est vrai que la compétence économique, la Shell des intercommunalités en la matière, l'hiver, rapporteur général l'bien indiqué : la répartition c'est aussi compliqué

qui ne perçoivent très peu qui espérait et puis qui perçoivent très peu donc en la matière je me relire et naturellement la position du rapporteur général au niveau de notre commission des finances, mais c'est vrai que je pense qu'il est important je dirais que, qu'on trouve des solutions à caractère financier ou autre voir peu des amendements d'appel parce que c'est là, c'est là qu'on voit que, il y a vraiment des peut-être pas par les dysfonctionnements, mais je dirais en la matière, je crois qu'il faut vraiment revoir un petit peu cette répartition on parle souvent de péréquation, bon je partage aussi, donc je me rallie à la position de notre commission des finances jour merci. Très bien, pas d'autres explications, donc je vais mettre aux voix. Ces 2 puisque l'on été retiré ces 2 amendements avec avis défavorable du gouvernement, Éric défavorable de la commission qui est pour.

Monsieur le président, le mini-cet amendement est exactement de la même inspiration. Donc que le précédent et je vois bien ce que vous allez me répondre et même la milice parmi les les arguments et aussi les arguments du rapporteur général, la rupture d'égalité avec une énergie qui serait notamment l'énergie nucléaire concernant l'hiver et évidemment un argument qui porte, c'est complètement évident qu'on est, par ses amendements en train de constituer une fiscalité de l'éolien, ce qui évidemment pas le pas l'objectif Le président m'aurait continué sa série de d'amendements en souhaitant une meilleure répartition de l'hiver éolien dans les EPCI à fiscalité professionnelle unique, donc je présume que vous allez me faire exactement la même réponse, mais je vais néanmoins l'attendre parce qu'on ne sait jamais, le pire n'est jamais certain. merci donc le 367 madame de Khomeiny. Oui, qui est bien défendu par ma collègue Nathalie Goulet, celui-ci est un peu différent dans la répartition me semble que le précédent demande 50 50 E répartition et dans cet amendement demande 30 pourcent pour les communes. Donc sur ces 2 amendements qui sont légèrement différents, monsieur le rapporteur général avis la commissions. Je disais tout à l'heure en introduction que lorsque les légifère, a été créé, je, je m'en souviens j'ai participé au débat il y a eu de très très nombreux débats sur la répartition des hivers entre les différentes collectivités, notamment entre les départements, le bloc communal et autres ces 2 amendements et réduisent ou ici pris la part départementale ça revient sur un équilibre qui avait été à l'époque, trouver qui est sans doute perfectible mais faut-il aujourd'hui alors que le département des finances, qui sont quand même fragilisée, alors qu'il y a un débat qui doit venir et auxquels on ne coupera pas sur la fiscalité et les ressources des différents des différents niveaux de collectivités et la perspective de la soupe sur le texte habitations durant ce débat absolument inéluctable est-ce que c'est le moment d'aller toucher un équilibre et de revenir au cours d'une loi de finances comme ça de manière par le biais d'un amendement sur des ressources, voilà pour les départements sera une paire de ressources, on a absolument pas capable d'en mesurer les conséquences par département, par quoi on compense cette perte de ressources, on n'en doute l'idée sans doute sympathique mais vous comprenez que la vie sera défavorable. L'avis du gouvernement. Donc même avis : il y a part du gouvernement, donc je vais mettre aux voix, il n'y a pas d'explication de vote Madame Goulet. retire, je retire tous les 2, j'ai bien compris et je pense que c'est à l'intérieur d'une meilleure péréquation à l'intérieur des intercommunalités ou ou avec un arrangement entre les collectivités elles-mêmes qu'on pourra éventuellement compenser ces ces pertes de recettes des premières collectivités qui ont été plus à l'avance sur les énergies renouvelables, je vous remercie.

Un amendement 246. Monsieur Gremillet. de sortir de de l'assiette d'imposition les passes à poissons et centrales hydroélectriques aujourd'hui dans le cas de la continuité écologique doivent réaliser des Pass à poissons qui d'ailleurs sont des investissements relativement lourds qui sont souvent cofinancé par l'État, cofinancé par les agences il serait quand même logique ou tout du mois elle n'apporte aucune plus- Value aucune production économique sont plutôt des contraintes à titre environnementale et il vous est proposé tout simplement de de sortir de taxe foncière, c'est pas ça passion. Alors un amendement. Identique de monsieur étaient plus de 154. Oui, il est rédigé, pas tout à fait de la même façon, je parlais plus d'installations hydroélectriques destinée à la préservation de la biodiversité de la continuité écologique mais je note que ce sont des Pass à poissons voilà, sinon, il est descendu. Très bien, ensuite, toujours en identique mais il ne sera pas défendu le 494 donc sur. 2 amendements, l'avis de la commission. l'avis de la commission. Ici, on ne vous surprendra pas, parce que parfois j'ai l'impression de, de, de, de, de me répéter, mais on a eu exactement ces mêmes amendements, l'autre jour en première partie du PLF, on considérait que je vais 18 îles qui proposé aboutir à une plus grande complexité il viendra évidemment réduire les recettes des collectivités territoriales et pour les raisons que j'avais exprimée en première partie, la commission est défavorable, ces amendements. Avis du gouvernement. Oui merci Michel, nous, nous considérons que la taxe foncière n'est pas un levier adéquat pour pour ce sujet et les exonérations de taxes sont chères doivent conserver un caractère extrêmement limité, donc nous sommes défavorables également. Bien, donc je vais mettre ces amendements, on voit qu'il n'y a pas de d'explications de vote. Avec des avis défavorables de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Abstentions. Donc ils ne sont pas adaptées.

Donc, cet amendement vise cette fois-ci à étendre les exonérations de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises, j'ai bien noté que j'allais sans doute avoir la même réplique du rapporteur général je je maintiens quand même cette fois-ci pour les installations de méthanisation et les sociétés de méthanisation agricole à toutes les installations et société méthanisation sur demande des collectivités territoriales cette exonération cette extension d'exonération pardon vise en effet à soutenir le développement de la filière et à valoriser la méthanisation des déchets non dangereux ou de manière ou de Bien, donc l'avis de la commission. facultative bien sûr et non compensées par l'État, cet arrêt rigueur de sa liberté locale et comme je suis pour la liberté, voilà, c'est un avis de sagesse, après tout, c'est le choix de la collectivité si elle décide de voter, c'est que générations alors suivi la pas de recettes, donc y a pas de raison de de le priver de cette faculté, donc la vie de sagesse sur cet amendement. Abbé du gouvernement. Oui le la vie est est défavorable. Le gouvernement considère d'autres types d'établissements que les établissements agricoles irait très au-delà de la situation actuelle en faveur des exploitants pour méthane ils aident leurs déchets dans une logique de proximité et de lutte contre la pollution agricole avec un Champ d'action aussi large, l'efficacité, d'autres mesures ni chiffré ni documenté comme sa pertinence paraissent problématiques, en effet, cette évolution conduirait à accorder une subvention à des entreprises industrielles, a priori, rentables et bénéficierait à certains géants du secteur, qui n'ont aucun besoin d'aide.

Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mischa collègues, j'ai pas une grande passion pour ce type de liberté pour les collectivités locales, je dois le dire

Pas d'autres explications de vote, donc je vais mettre aux voix cet amendement avec un avis de sagesse de la Commission, un avis défavorable du gouvernement qui est pour.

Le 613 propose d'exonérer diffère les stations de transfert d'énergie par pompage, ce qui représente un montant de 13 millions d'euros par an, pourquoi ça serait en effet un signal fort pour la mise en 9 des objectifs de développement du stockage objectifs et moyens de la politique énergétique française tels qu'inscrits dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, avec un objectif de création de un à 2 gigawatts supplémentaires de Step entre 2025 et 2030.

Et pour y arriver. Ensuite, nouvel amendement toujours sur le même article. Le 250 Monsieur pu. Alors cette fois-ci il s'agit de l'article 265 du code des douanes qui prévoit la CGT cela sujet tisse ment à la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant combustibles cet amendement propose d'inscrire à cet article le principe d'une composante carbone des taxe intérieure de consommation assis sur le seul contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis, cette mesure permettrait donc d'exclure la composante carbone les produits issues de la biomasse.

Bon. Première partie : la loi de finances il y a une raison pour laquelle cette amendement, on ne peut pas être accepté, c'est tout simplement parce que il ne modifie pas les tarifs, donc il était inopérant, il n'apporte aucune conséquence juridique et de ce fait c'est pas vraiment un amendement de loi de finances était un plutôt une pétition de principe mais sans modification de tarif, voilà la loi, je m'en un sens de pas simplement poser des tarifs des principes mais également tirer les conséquences juridiques, ce qui ne fait pas d'amendement, c'est donc un avis défavorable. Et du gouvernement. Défavorable. Défavorable. Pas d'explication de vote donc je mets aux voix avec un avis 2 avis défavorables de la Commission et du gouvernement qui est pour.

C'est le dernier pour cette série. Non, non pas que vous médias usé mais cette amende, or dans le vise à rétablir la taxe sur les gaz HFC qui avait été proposé en commission du développement durable, sur la première partie du PLF puis retiré propose donc une clarification par rapport au précédent texte étudié en commission en explicitant mieux la modification apportée à l'article 266 des siestes du code des douanes je ne développe pas plus avant. Avis de la commission, un monsieur de Montgolfier. Défavorable. Favorable à l'du gouvernement. Défavorable. Défavorable, donc pas d'explication de vote je mets aux voix qui est pour.

Merci monsieur le président je présente cet amendement non de notre collègue Berry de bas et du groupe socialiste sur. Les les transports qui représente un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre et son nom grandement responsable de la pollution de l'air sous la forme de gaz et particules fines dont on connaît les effets désastreux sur la santé et dont le coût pour la société est énorme, la pollution de l'air et la cause chaque année de milliers de décès prématurés, plus de 480000 personnes au sein de l'Union européenne en 2014, il est donc urgent de s'attaquer à ce fléau et le parc automobile français très ancien, composée de véhicules polluants voire très polluant et contribue grandement à cette pollution. On ne dénombre en effet pas moins de 3 millions de véhicules essence datant d'avant 97 et de 7 millions de véhicules diésel datant d'avant 2006, le ministre de la transition écologique et solidaire, a souhaité en faire un des enjeux primordiaux de son plan climat, avec l'objectif d'atteindre la fin de la vente de véhicules thermiques d'ici 2040, dans cette optique, certains dispositifs sont prévues afin de favoriser le remplacement des véhicules thermiques polluantes augmenter la taxe carbone, faire converger la fiscalité du gazole et celle de l'essence sont par exemple des facteurs incitatifs à la réduction de la consommation de produits à fort contenu carbone mais pour incitative, qu'elle soit cette fiscalité écologique n'en est pas moins régressive et risque d'impacter fortement les ménages aux revenus les plus modestes qui ne pourront, faute de moyens financiers suffisants remplacer leur véhicule polluant par un véhicule propre, c'est donc la double peine, si le gouvernement a prévu des dispositifs d'aide et d'accompagnement, comme la prime à la conversion de 2000 euros pour les ménages non imposables. On peut craindre que ces aides ne soient pas suffisantes pour leur permettent de remplacer leurs véhicules anciens par un véhicule propre, cet amendement vise à compléter ce 1er dispositif car il faut réussir de manière massive à mettre au rebut les véhicules polluants et cela suppose des aides conséquentes et un accompagnement conséquent des ménages à revenus modestes, donc cet amendement très concrètement, propose la mise en place de prêts à taux 0 pour permettre à ces ménages d'acheter un véhicule 9 ou d'occasion, propres, en contrepartie de la mise au rebut du véhicule polluant dont ils sont propriétaires donc il complèterait ce dispositif de manière nous sommes très opportune la prime de conversion. Mise en oeuvre et de ne pas pénaliser les foyers à revenus modestes, en favorisant l'accélération de la mise à la casse des véhicules polluants, je vous remercie. On ne peut que partager les objectifs de l'auteur de l'amendement d'accélérer la conversion, les disparitions des véhicules les plus polluants et c'est d'ailleurs l'objectif de la prime à la perversion avec pour le le garnement je pense des objectifs qui sont très ambitieux, seront-ils atteints, c'est une vraie question : quand on regarde très concrètement, le nombre de de et la sous-consommation des crédits, il sera pas tout à fait, tout à fait évident, c'était pas ça, ce pas encore assuré qu'on sera capable de distribuer 100000 primes comme l'ambitionne le garnement

donc, faut-il le redire dispositif avec un nouveau dispositif de prêt à taux 0, sachant que très souvent, les constructeurs automobiles d'ailleurs faut des opérations promotionnelles sur le crédit

Merci à vie du gouvernement Madame le Ministre. Oui merci monsieur le président. Je voudrais exprimer donc le le le le soutien du gouvernement à l'effort, il y a la conversion des des véhicules polluants. On a rappelé la prime à la conversion qui qui renforcée en 2018 le bonus électrique qui est maintenu à un niveau élevé le barème de taxe sur les véhicules de société qui sera modifiée en 2018 en faveur des véhicules les moins émetteurs de CO2 et les moins polluants polluants, le plafond de déductibilité de l'amortissement qui a été modifié en 2017 en faveur des véhicules les moins émetteurs de CO2 et sera maintenue en 2018 donc toutes ces mesures vont dans le bon sens, en revanche, le gouvernement ne peut soutenir votre proposition d'élargir le mécanisme du prêt à taux 0. un investissement véhicule, ceci n'est pas son objet et donc nous sommes défavorables à votre amendement merci.

La forêt formidable puits de carbone, les estimations indiquent que la forêt française en stock fait environ 1,1 milliard de tonnes, soit 80 tonnes avec, il convient d'étudier les mécanismes financiers à mettre en oeuvre pour compenser l'absence de ressources générées par les forêts non exploitées et participer ainsi au financement des coûts de leur gestion, surveillance et préservation les collectivités en assume une grande part, soit directement sur leur participation auprès des organismes délégataires comme l'ONF ou les parcs naturels, ces compensations pourraient également venir aider à valoriser les filières d'agroforesterie faiblement émettrice de carbone, voire de stockage à long terme de carbone comme le bois d'oeuvre, par exemple, à titre d'exemple conomie sociales et environnementales dans son rapport de 2012 sur la valorisation de la forêt française préconisait que la France se dote de moyens compensatoires pour répondre aux défis auxquels est confrontée la forêt tropicale guyanaise, en effet, concernant l'accessibilité au crédit carbone la France pays inscrits à l'annexe, ça n'est pas éligible aux mécanismes Red plus alors qu'elle est un des pays financeurs de ce mécanisme à disposer d'un couvert forestier tropical important le puits de carbone de la forêt amazonienne de Guyane, laquelle a une superficie de 7,5 millions d'hectares séquestre près de 15 millions de tonnes de CO2 par an, contribuant ainsi à hauteur de 20,7 pourcent à la fin, international de CO2.

Merci Monsieur le Président, la ville où gouvernement et une demande de. Il s'agirait documenté, l'absence de ressources générées par les forêts non exploitées et ainsi de participer au financement des couleurs gestion surveillance et préservation la production d'untel rapport ne paraît pas justifié, s'agissant d'un sujet qui ne doit pas être abordé sous le seul angle restrictif des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales. Ainsi, sur cette demande de rapport parce que vu le nombre d'interdiction qui frappe l'exploitation des ressources naturelles, Guyane, la prise en considération de ce puits de carbone, une excellente peu partie quand sait que l'exploitation de d'hydrocarbure ne peuvent pas être possible en Guyane française, alors qu'elle est dans tous les pays voisins, qu'il y a beaucoup de d'interdiction en matière d'exploitation minière que la forêt primaire également et mise sous cloche, il est quand même normal que la Guyane à Parme, juste retour de ce puits de carbone. Est-ce qu'il y a des explications de vote, je vais mettre aux voix avec de demandes de retrait de la Commission et du gouvernement, vous ne retirez pas Monsieur passion non vous maintenez qui est, qui est favorable. Défavorable. Abstentions. Donc l'amendement n'est pas adopté

après l'article. 39 d6 donc de nouveaux amendements pour un article additionnel Madame il n'est pas soutenu. Donc je mets on voit ensuite l'article 39 indécise. C'est pour dire on. Abstention donc il est adopté, on attaque l'article 10 l'article 40, pardon, l'article 40

Monsieur Bocquet. Oui, merci Monsieur le Président, effectivement, au moins 149 on a l'impression que le versement nous propose quelque part de couper la France en 2 du point de vue de la politique d'accession sociale à la propriété d'un côté, plus de 33000 communes, c'est l'immense majorité d'entre elles, mais aussi une bonne part des villes préfectures tout de nos départements où le PTZ ne serait plus mobilisés que sur le marché de l'ancien. c'est évidemment l'activité du bâtiment risque de grue gravement subir les conséquences de ses choix, ne serait-ce que parce que, pour ne donner qu'un exemple de réserver l'Opinel cojones tendue, on en a parlé tout à l'heure, conduit à rémunérer la rente foncière en première instance et a tiré sur les prix de la construction en elle-même, avec ce que cela implique et notamment parfois le recours à des entreprises qui, en matière sociale ou d'organisation du travail ont dépassé depuis longtemps leur quota de droit à l'erreur, selon l'appellation du jour, il serait tout de même dommage que la priorisation définie par l'article 40 conduisent à mettre en question le dispositif même d'accession à la propriété et que l'équation budgétaire ne se résolvent par le recours au travail précaire et ou dissimulé, n'oublions pas que les accédants du prêt à taux 0, malgré ce que l'on peut dire du plafond des revenus constituent une population aux caractéristiques sociales très proche de la population des cités de logements locatifs HLM merci. Merci donc l'amendement suivant le 441 n'est pas défendu. Le 596 Madame Lienemann. Oui ben c'est un amendement qui va dans le même sens, qui vise à garder le PTZ sur l'ensemble du territoire national pour une raison simple, c'est que les seuls outils de l'accession sociale à la propriété sont d'abord le PTZ et d'autre part, le PS et là qui va encore pour les catégories un peu plus modeste que la moyenne du PTZ alors est-ce qu'on veut une France où on dit à nos concitoyens qu'habitent en zone B2 et C : circulez, il y a rien à voir, il y a plus de politique publique pour vous.

que réduire le PTZ comme le soleil prévue, va faire une hémorragie considérable l'sur ces territoires dans l'accession sociale à la propriété, moi je crois que l'accession sociale à propriété était un des éléments du parcours résidentiel qui permet aux catégories modestes et populaires, au

Ethan est un outil pour permettre des constructions relativement raisonnables sur ces secteurs et donc nous défendons l'idée qu'il faut maintenir ces PTZ dans la durée et sur l'ensemble du territoire national. Merci donc l'amendement suivant Monsieur Bocquet ou monsieur Ouzoulias. Oui, j'enfonce le clou, parce que sur ce sujet, pour une fois on chasse en meute en apportant quelques quelques chiffres complémentaires pour vous dire simplement que les zones C et B 2 c'est 33613 communes, c'est pas un petit chiffre et aujourd'hui, ça représente 60 pourcent des prêts à taux 0, donc si on enlève ces 2 zones tout le dispositif et vidé de son sens et c'est la disparition du prêt à taux 0 merci. Eh bien, le 597 Madame Lienemann. Non, c'est un amendement de repli si par malheur mais je crois quand même que dans beaucoup de rang du Sénat, on est très attentif à l'accession sociale dans l'ensemble du territoire et que les élus de des territoires, notamment ruraux, mais aussi des villes moyennes et même de la grande couronne de nos métropoles voit bien à quel point c'est nécessaire si telle n'était pas le cas, je propose qu'on maintienne le PTZ temps plein pour accompagner la procédure de paix, c'est là, je vous rappelle que c'est la location accession que cette procédure touche des catégories très modestes et c'est justement dans ces zones que les catégories modestes peuvent accéder à la populaire. à la à la. Propriété et, par ailleurs, je voudrais insister sur le fait que concentrer le PTZ en zone et en zone A B 1 B 2 B I c'est accompagner la hausse des prix, ça ne fera absolument pas à une amélioration de la solvabilisation des accidents génie rien contre, mais je dis que par rapport à ça, on va avoir un frein considérable dans l'accession sociale à la propriété. Bien, merci pour le 704 maintenant Madame de remédier. Oui, merci Monsieur le Président, écoutez, je crois que nous sommes tous d'accord sur ça, donc nous insistons pas le présent amendement propose donc de maintenir une quotité près identique sur l'ensemble du territoire. Merci, toujours dans la discussion commune le 548 rectifier Monsieur Delcros.

qui veulent accéder à la propriété dans un cas, on va le réduire, hé bien écoutez vous construisez dans telle zone ou dans telle ville et je suis d'accord à ce qui interdit sur le prix du foncier est à l'heure par Marie-Noëlle, vous allez pouvoir financer 40 pourcent de votre opération de votre construction mais ce couple qui veut construire en milieu rural parce que son travail est là

dans laquelle il y a pas beaucoup temps beaucoup de constructions mais on a besoin justement au au nom de l'équilibre des territoires et de la répartition de la population sur l'ensemble du territoire national, on a besoin d'envoyer des signes positifs et avoir cette mesure discriminatoire pour les jeunes, pour les familles, pour les primo-accédants qui, souvent, je suis d'accord sont plutôt des familles qui n'ont pas des revenus considérables, je, je trouve que c'est dommage, donc, un vrai sujet, on apporte une mauvaise réponse, on a des solutions, s'il faut réduire la dépense, y compris sur ce gel, il y a des solutions qui arriveront pas qui seront pas discriminatoire vis-à-vis des jeunes et des primo-accédants. Très bien, merci, donc, sur ces amendements, discussions communes l'avis de la commission du rapporteur général. La commission des finances n'a pas souhaité modifier l'article 40 puisque nous considérons que le zonage pour le 9 et pour l'ancien, et plutôt pertinent recentrer le 9 sur les zones tendues, là il y a besoin de plus de production de logements, ça nous semble utile évidemment avoir le sur les zones, au contraire, détendu, là où le besoin de rénovation, le, le PDG d'sur l'ancien, ça nous semble également pertinent et avec les dispositifs transitoires de de permettant de logique bénéfice du dispositif, appelle qu'on est parvenu à un équilibre, tous les autres si on adoptait l'un ou l'autre de ces amendements, évidemment, il y aurait tout de suite, ils portent bien leur nom et s'appelle Artis 40 ils aggraveraient les charges d'eau qui contribuera évidemment à et augmenter la dépense fiscale qui est déjà élevé, c'est presque un milliard d'euros, et donc la Commission continue des avancées à l'Assemblée nationale sur cet article 40 a souhaité en rester là et c'est la raison de la, de l'avis défavorable de demandes de retrait sur cette série d'amendements d'extension de maintien du PTZ de suppression de conditions de zonage ou d'application de, de, de, de différentes quotité pas déterminer le montant du PDS, sans condition de localisation, donc tout ça m'ennuie, on va dans le sens, une somme qui on est parvenu à un équilibre et toute extension évidemment auraient des conséquences budgétaires qui nous paraissent incompatibles avec l'objectif de maîtrise de la dépense fiscale donc avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, donc même dans la vie du gouvernement Madame la ministre. Oui, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Oui, merci Monsieur le Président, le le gouvernement est défavorable à l'ensemble de ces amendements qui conduirait à significative significativement l'équilibre de ce qui a été proposée en terme de recentrage du PTZ donc on on cherche ici la rationalisation, une meilleure efficacité et on se trouve donc dans un dispositif qui est déjà très coûteuse tout élargissement généralisation. Oui conduirait en effet à déséquilibrer ce ce budget de quelques centaines de millions. D'euros

C, on veut plus de HLM, on nous a expliqué hier, il fallait mais tout l'argent dans les secteurs où soi-disant dans les zones tendues fallait recentrer, on veut pas d'accession sociale à la propriété il faut le dire, et après vous viendrez pas pleurer de voir passer les extrêmes les populismes s'installer sur ces territoires, vous ne donnez aucune perspective aux jeunes qui vivent et à l'ensemble des gens qui espère avoir un peu de promotion sociale, deuxièmement, vous nous dites c'est coûteux, alors oui, 100 millions d'euros, je vous rappelle que, quand vous avez doublé l'Avantage aux stock-options à l'Assemblée nationale, ces 120 millions d'euros. Où est l'intérêt national. Je ne crois pas que le doublement des stock-options à plus d'impact économique sans parler de son impact social que les 100 millions sur le PTZ troisièmement si vous voulez recentrer le PTZ, il faut le recentrer par rapport aux ressources. Et pas par rapport au territoire et que par ailleurs, c'est d'ailleurs pourquoi je plaide pour qu'à minima, si nous ne gagnons pas sur le PTZ sur l'ensemble du secteur B 2 et c'est au moins pour le PS, et là, donc je vous rappelle qu'il y en a que 10000 par an.

Maintenant, il y a plus rien dans toute une partie du territoire, alors moi je n'ai jamais été pour le tous propriétaires : je suis pour que l'accès sur ceci à la propriété, puisse être maintenue, comme un des piliers des politiques complémentaire au locatif social. Merci, la parole monsieur Delcros. Oui les les réponses faites tant par le rapporteur général que par Madame la Ministre, laissent à penser, à tort, que tous ces amendements visent à accroître

quelque que soient les territoires sur lesquels elle s'installer quelque soit les territoires sur lesquels j'ai envie de construire parce qu'ils ont choisi d'habiter là ou parce qu'ils ont leur travail, on les traite de la même façon de manière équitable sinon mais vers quelle France on va vers quelle France en bas avec ce type de disposition. Merci, ce que j'ai d'autres explications de vote sur ces amendements, pas d'autre explication de vote donc je on voit successivement le 649 donc avis défavorable, bien entendu, de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est content.

Adopté l'amendement 649 est adopté. Le 596 avec avis défavorable de la commune. Non, il tombait effectivement, pardon, c'est le même. Ensuite, le 641 tombes aussi. Non 597 présenté par Madame Lienemann voter. Donc, sur 597 qui est favorable, inquiet pour.

Donc, le 704 maintenant qui était présentées donc par Madame de Romilly, celle qui l'a présentée avec avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Sur les 704 qui est pour.

Donc je 548 est adopté. J'aimais on voit l'article 40. Pas d'explication de vote.

et au regard des objectifs partagés tant par les élus de terrain que les institutions le monde HLM et les opérateurs déterminant, parfois même le seul en territoire détendu, on observe que le prêt à l'accession sociale a permis de financer près de 73000 opérations en 2016 65 réalisé dans l'ancien et 60 pourcent en zone rurale, ces chiffres confirment qu'il s'agit d'un bon outil pour intervenir dans les centres notre amendement propose donc de permettre aux conseils départementaux qui le souhaitent d'exonérer de droits d'enregistrement, les ventes de logements qui se réalise dans la cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété en centre bourg, c'est-à-dire liées aux prêts d'accession sociale, il répond à l'objectif du plan villes moyennes qui a été lancé par le gouvernement en février 2010 et qui doit être ah oui, qui mais qui a été déjà annoncée par le ministre, mais ça, et donc nous pensons que cette mesure n'est est une liberté donnée aux collectivités est un outil qui leur permet d'accompagner la revitalisation de leurs centres bourgs et des villes moyennes.

de sa je crois supprimer la part départementale des droits de mutation, ce que pour autant ce sera incitatif donc tout, c'était plutôt une demande de retrait une interrogation face à l'efficacité avait été l'outil de suppression d'oedèmes L'avis du gouvernement n'administre. Même avis. Donc sur cette demande de retrait Madame Lienemann. Oui, hé ben oui, c'est un bon outil pour une raison simple, c'est qu'il y a déjà des opérations qui sont discutées avec les départements dans certaines zones rurales ou de villes moyennes et qu'aujourd'hui on n'a absolument aucun opérationnel, alors évidemment les départements vont pas aller se précipiter à le faire n'importe comment, sous n'importe quelles conditions puisque ça leur les prive de ressources mais j'entends bien Monsieur le le rapporteur, que tout à l'heure, vous vous disiez qu'il fallait donner des libertés aux collectivités, c'est à elle de faire l'arbitrage s'il considère que l'accession sociale dans le centre bourg où les centres villes moyennes est un outil de leur développement, moi je ne vois pas pourquoi on s'y oppose, je le dis d'autant plus que on ne revitalise centre ancien que par un mixte entre l'accession sociale et du locatif, une des faiblesses de nos opérations de réhabilitation à travers les opérations Anna ont été de tellement concentrés sur simplement du locatif à caractère social toujours utile, mais qui ne suffit pas à recréer une mixité attractif pour les centres villes moyennes et debout.

et que ce soit le bon moment pour les départements d'par des recettes néanmoins j'entends ce que vous dites et pas au principe de liberté chérie par tous, ici, hé bien je me remets à la sagesse du Sénat.

notre position sur le CIC, le hier, je connais la réponse de notre rapporteur général à la réponse du gouvernement, donc je vais pas développer, mais simplement une information quand même, comme chacun le sait, nous avons vu s'engager ces derniers temps, ces dernières années un processus de baisse du taux facial de l'impôt sur les sociétés qui pose d'incontestables question parce que la réalité de ce que perçoit l'état en bout de course, n'a rien à voir avec le taux affiché à l'origine, comment, en effet, avec un PIB marchand de 2200 milliards d'euros à peu près arriverons-nous à un impôt société brute de 57 milliards d'euros, soit 2,5 pourcent environ, ce qui est la moyenne de prélèvements apparent, l'Union européenne, rappelons-le au passage, pour un rendement Net de 28,4 milliards d'euros une fois déduit le CICE Le crédit d'impôt recherche quelques autres également, sans oublier le report en arrière de déficit antérieur, voilà, c'est dire que notre impôt société représentent environ effectivement 1,3 pourcent du produit intérieur brut, voilà la réalité de certains chiffres merci.

très concrètement, vous savez, évidemment que la réponse sera défavorable alors dans un grand quotidien économique du matin qui me passe à des collègues, il y a un titre à la pression fiscale en France est la plus élevée de l'Union européenne et la France se situe un ratio de recettes fiscales PIB en 2016 pourcent devant le Danemark, la Suède, l'Italie et bien sûr la moyenne de la zone Euro, donc nous sommes le seul pays qui a la pression fiscale et à des taux d'imposition sur les sociétés par vous savez les plus élevés d'Europe la majorité sénatoriale n'approuvent pas tous la politique fiscale gouvernement mais un art je m'elle prouvé la trajectoire de baisse de la Poste société il serait catastrophique, dit revenir avis très défavorables. Merci avait du gouvernement. Défavorable, pas d'explication de vote. Je donc je mets au voile 477 qui est pour. Qui est contre, abstention, il n'est pas adopté, je mets au voilà requis que 41 pour l'article 41 qui est pour. C'est con. Abstention : l'article 41 est adopté. Donc article additionnel après l'article 41 propositions, en tout cas Madame couler le sang, 68 rectifier. Oui, Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, alors là, nous abordons un sujet qui fâche, qui la fiscalité numérique, alors on va me dire qu'il y a un rapport, on va me dire qu'il y a un texte qui, arrivant même dire que c'est de la compétence de l'Union européenne, on va me dire. Que le mini s'en occupe néanmoins puisque nous sommes dans le cas de la loi de finances et que c'est quand même un exercice tout à fait habilités pour pour pouvoir présenter des propositions, je vous propose cette cette proposition sur un régime d'imposition de certains services fournis par voie électronique, cet amendement instaure une obligation de déclaration pour les entreprises du numérique qui existe, qui exercent leurs activités en France et qui ont leur siège dans un autre État de l'Union européenne, cet amendement soutient par ailleurs la création d'une taxation sur la publicité en ligne, je vous rappelle que cette disposition avait été adoptée par l'article 27 de la loi du 29 décembre 2010, loi de finance donc pour 2011 avant d'être abrogée par l'article 19 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative, donc il y a eu une brève période de lucidité, où on a appliqué cette disposition, puis elle a disparu de façon magique, moi je crois qu'il est temps de de donner, de donner un signal, on travaille tout ce nouveau réfléchissons sur une taxation des GAFA on sait tous que c'est extrêmement compliqué, mais là, en même temps, il s'agit d'une déclaration et je pense que c'est c'est un 1er pas vers une possibilité d'encadrer une taxation sur sur des activités qui échappent complètement à l'impôt, c'est c'est l'objet de cet amendement, qui est d'ailleurs un amendement qui a été repris par l'ensemble du groupe de l'Union centriste en aura plusieurs, de ce genre dans le cours des débats j'observe dans les 33 secondes qui me restent, que nous avons adopté 210 amendements depuis ce matin, qu'on pourrait bien passer un peu de temps sur la fiscalité du numérique. Madame Ray, monsieur le rapporteur général, avis de la commission. Grâce à Génération Nathalie Goulet, la commission des finances à laquelle elle est partie et a passé beaucoup de temps, il passera beaucoup de temps, c'est un sujet qui, concrètement, est un sujet pour nous extrêmement important, au-delà de la publicité en ligne, simplement, la tension est très louable mais cette amendement, il ne semble manquer totalement sa cible, moi je prends 2 2 exemples très basique, la régie publicitaire est en France qui est ce qui va se passer, elle va répercuter sur les annonceurs, le prix de la taxe évidemment et ça ne changera strictement rien à la situation se sera les annonceurs qui seront les perdants et en aucun cas le l'annonceur et autres et la taxation des profits du numérique, c'est une autre question sujet situation le régie publicitaire se délocalise à l'étranger et dans ce cas-là, évidemment, on peut l'envoyer tous les papiers bleus qu'elle veut, elle ne paiera jamais la taxe publicité en ligne il y a 1er territorialité de l'impôt donc Dog fait avoir une taxe sur la publicité tendu d'une idée extrêmement sympathique, ce qu'il faut taxer ceux non pas la publicité, c'est les bénéfices des multinationales et entreprises du Gard qui vivent de la publicité en ligne, mais en aucun cas les régies publicitaires, soit en France répercuteront relate que la taxe soit installé étrangers la paieront pas, donc ça me, raison pour laquelle ça me semble pour le coup, être contreproductif et le seul effet sans doute de cette amendement s'il était voté, ça serait cap une régie publicitaire en France et sa mère, et tout à l'étranger, et ce serait sans doute le risque donc c'est avis défavorable mais je rationaliser Goulet, nous aurons un retrait sur les sujets du numérique en a beaucoup, beaucoup. Merci l'avis du gouvernement, mais la ministre. et continuera à poursuivre le ministre Bruno Le Maire s'est engagé à le porter et à et fortement au niveau européen et c'est vraiment au niveau européen qu'on pourra trouver des solutions satisfaisantes et opérante sur ce type de sujet en l'espèce par son assiette limiter la taxe proposée s'ajoute à un ensemble de petites taxes déjà existantes en France, sans apporter d'innovation quant à la mise en compte la prise en compte de la création de valeurs générées par les acteurs du numérique, compte tenu du seuil d'imposition établi à 20 millions d'euros pour les sommes versées par les annonceurs, régies publicitaires, cette taxe ne peut qu'avoir rendement très limitée, elle n'apporte donc aucune réponse à la taxation des grandes entreprises des grands acteurs internationaux du numérique et donc je suggère le retrait de cet amendement.

qui vise à considérer que sont établis en France des établissements quand il dépasse en millions de chiffre d'affaires, on taxe pas le chiffre d'affaires, mais on le reconnaît comme établi en France à partir du moment où il y a 100 millions et là on applique notre législation normale, ce que font les Anglais, en plus, ils mettent des et des amendes, mais ce serait pas constitutionnel, chez nous, donc on aura ce débat, j'espère que le Sénat renouvellera son son vote, on a travaillé la compétence, la compatibilité avec les normes OCDE européenne l'épreuve les Anglais avant le Brexit, l'avait fait mais, Madame la Ministre, voyez, on n'arrive plus à croire ce discours.

on attend quoi, on peut, on doit agir en Europe, moi je reconnais au gouvernement sa volonté de mobiliser l'Europe, j'observe que c'est pas de mal avec on a une majorité jeudi utilisons toutes les marges de manoeuvres, la France possède pour utiliser au mieux ses marges demain 9 pour taxer davantage les multinationales, les GAFA et donc je pense madame voulait en effet votre amendement n'a peut-être pas une pertinence technique en la matière, j'espère que vous retiendrez celui que nous avions déjà voté mais par signal politique de solidarité avec vous pour ce débat et lieu de manière permanente et notamment dans la navette, j'ai pour ma part je voterai votre amendement. Merci, Monsieur Bocquet. par la volonté qui transparaît dans la composition de la liste noire des paradis fiscaux publiée mardi dernier, permettez-moi de douter de cette volonté farouche d'éradiquer le phénomène, c'est une plaisanterie, son nom.

donc je mets aux voix s'il n'y a pas d'explication de vote l'amendement de Madame Goulet, qui n'est pas retiré puisqu'il y avait une demande de retrait maintenu donc sur cet amendement, qui est pour.

l'amendement est adopté, Alors, après l'article 41 l'amendement 164 et qui fit Madame Nathalie Goulet. Oui, Monsieur le Président, alors là nous sommes dans un dans un amendement qui est la transe. Philippe Sion d'une proposition issue des travaux de la commission sénatoriale que nous avions eues sur l'évasion fiscale, donc ça fait plusieurs fois qu'on remet cette disposition sur le tapis à chaque loi de finances à Châtelet à chaque loi de finances rectificative chaque fois qu'on a un débat sur la politique fiscale, nous remettons le métier l'ouvrage sur le métier, donc cet amendement concourant à l'amélioration de la transparence financière internationale, il entend accorder la publicité nécessaire aux éléments constitutifs de la stratégie globale des entreprises engagées dans une compétition internationale en parfaite adéquation avec les recommandations de l'OCDE, qui ont d'ailleurs bien progressé depuis nos commissions d'enquête avec les bêtes, et de ce point de vue là on a quand même beaucoup avancé, il fournit ainsi un instrument précieux dans la lutte contre la fraude fiscale et sociale, il s'agit en fait pour les sociétés comme côté et celle qui a la date de clôture du bilan dépasse les limites chiffrées qui figure dans l'amendement de publier des informations sur leur implantation incluse dans le périmètre de consolidation de chaque État ou territoire au plus tard dans les 6 mois de la clôture de l'exercice, donc il s'agit d'un élément de transparence, je sais qu'on va commencer à dire que il y a le secret des affaires, etc, mais on est quand même dans les sujets dans les sujets de consolidation et on sait très bien comment ça se passe la commission d'enquête, qui a rendu son rapport, une fois en 2011 : une fois en 2012 ou 2013 il y a eu les Panama Papers, il y a les Paradise par tous les jours, nous sommes envahis de de scandale en ce qui n'est pas Rabat et ce n'est pas en ce qui concerne ses sujets et il y a fort à parier que, sans les Paradise Papers la liste la la liste de l'Union européenne ne serait jamais sorti il était pas du tout dans les tuyaux, l'Union européenne de ressortir une liste des territoires non-coopératifs, c'est simplement le scandale des Paradise Papers, qui a contraint l'Union européenne à revenir sur une liste des territoires non-coopératifs, donc voilà l'objet de cet amendement. Merci donc lundi de la commission.

effectivement la transparence, l'une des armes, à mon avis pour avancer enfin sur ce problème, nous ne sommes pas encore, loin s'en faut, donc nous sommes tout à fait favorable à ce que de nombreuses ONG portent depuis de nombreuses années sur le reporting pays par pays, pardon pour ce jargon un peu technique, et voilà qu'on en sache un peu plus son exige et c'est normal dans la République, la transparence des parlementaires et des élus, nous demandons, celle des grands groupes aussi. Très bien, donc, sur ces amendements la de la commission. Réussira dans cette matière très complexe que dans un cadre international très concrètement les les 2 cartes, si vous le savez, c'est le CDE c'est le la Commission européenne, on peut dire ce qu'on veut des listes noires, vertes rose et grise ou ce qu'on veut

c'est une avancée, ça été introduit l'échange automatique d'informations, ça a été également conclu par la France en janvier 2016 et il y a désormais 65 États qui ont en font partie et vous avez également bien sûr en tête le projet directive par la Commission européenne qui était et du 12 avril 2000,

on arriver aujourd'hui à des avancées considérables, ce n'est pas encore parfaite type il y a encore des, des, des discussions, je rappelle que la dans le projet, directive européenne de seuil serait à 750 millions d'euros, avoir en France un seuil de 100 millions d'euros différent du du seuil du secrétaire national serait extrêmement risqué et ne pèse au final de ces entreprises françaises donc encore une fois, vouloir faire les choses seul au risque d'être les plus vertueux, l'Europe ne produira aucun effet, par contre, s'engager dans le processus,

Madame Lienemann. J'entends bien l'argument de notre rapporteur, on a déjà eu ce débat, rappelez-vous, au moment des banques ou on nous expliquait que la France ne pouvait pas voter le reporting public rappelez-vous pour les banques parce qu'il fallait attend que l'Union européenne ne fasse en entre- temps. D'autres pays de l'Union européenne l'avait fait L Union européenne elle-même a fini par le voter parce que la crise bancaire étant tellement visible que c'était difficilement contournable, j'attire votre attention sur le fait que notre constitution parce que il y a eu un débat sur le reporting public avec le précédent gouvernement, on avait voté l'Assemblée avait voté le ce reporting public qui a été considérée comme anticonstitutionnelle et il ne pourrait redevenir constitutionnel en France que parce que ce serait votée au niveau européen en cela notre rapporteur a raison pour que la directive sur le reporting public devienne acceptable en France regarde notre constitution, d'après le Conseil constitutionnel, ça ne peut être que par la mesure européenne puisque vous savez que le droit européen s'impose au droit français, au passage, je considère que c'est révélateur d'une faiblesse constitutionnelle de notre pays, quand on a la transparence due au citoyen et aux organes publics pour autant, je pense qu'il faut qu'on donne un signe politique, notamment au Parlement européen aux instances européennes, dire que la France engage de toutes ses forces pour ce reporting public moi j'aurais souhaité qu'on puisse être allant tout seul comme certains pays l'ont été au moment des banques, on votera donc cet amendement et on souhaite qu'il y a une mobilisation générale de notre pays pour que ça aille maintenant très vite parce que j'ai cru comprendre qu'il avait encore bien des résistances pour faire avaliser cette directive.

de progrès, ces 3 dernières années que que les que les 10 derniers c'était évident qu'on a fait des progrès et c'est aussi évident qu'il faut donner des signaux, c'est la raison pour laquelle on maintient cet amendement. Merci, si j'ai pas d'autre explication de vote j'aime est-ce. Ces amendements voit d'abord qui sont pas tout à fait identique donc le 164 avec avis défavorable de la commission avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre.

compte-tenu de l'avancement de nos travaux, qui ce matin et cet après-midi nous ont permis d'avancer de façon quand même substantiel et de la disponibilité quelques créneaux travailler lundi, je pense que nous pourrions envisager l'arrêter vers 18 heures 30 sans nous réunir ni ce soir ni pendant le week-end de reprendre lundi à 10 heures si nous travaillons encore une heure de façon à peu près appliqué Astra 2 lors d'une centaine d'amendements, lundi, ce qui est tout à fait improbable.

dont acte, c'est on va fonctionner suivant ce régime c'est-à-dire que jusque vers 18 heures 30 on finira sur un chapitre, et ensuite une reprise des travaux lundi en en vous remerciant de cette proposition. Nous continuons donc après l'article 41 bis, j'ai des amendements.

par le Sénat de son amendement 649 donc ça va peut-être nous porter chance, voilà, on va donc parler du Rhône, vous l'imaginez bien, c'est son département alors que nous dit ce fameux article 41 bis déposé en catimini à l'Assemblée nationale par les députés de la majorité du Rhône au prétexte que la métropole de Lyon est une collectivité à statut particulier qui exerce des compétences d'élargie, cet article a pour conséquence d'exclure du Champ de l'article 89 de la loi de finances pour 2016, le territoire de la métropole de Lyon, en d'autres termes, cet article permet à la métropole lyonnaise de bénéficier de ressources dynamiques supplémentaires en modifiant la quote-part de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises la c'est VAE cela permet ainsi tout bonnement à cette métropole d'être exempté de versement de 25 pourcent de la CVE à la région Auvergne-Rhône-Alpes que cette dernière doit percevoir en 2018 au titre de la compensation du transfert de compétences, comme le prévoit la loi nôtre une disposition, lui permettant ainsi d'augmenter ses ressources fiscales, le tout bien sûr au détriment de la région Auvergne-Rhône-Alpes en créant un principe d'exception ainsi le présent amendement vise à rétablir l'égalité républicaine, les territoires et les collectivités, mais entend également éviter la création de métropoles à 2 vitesses. Merci donc en discussion commune, j'ai 313 monsieur Gremillet. Oui, merci Monsieur le président, mesdames, Nice Monsieur rapporteur général, chers collègues, l'amendement revient sur les conditions de financement prévu dans la loi, notre du transfert aux régions de la compétence départementale des transports non urbains, a instauré un traitement spécial unique en France pour la seule métropole de Lyon, le financement de cette compétence départementale vers les régions est fondée sur un transfert de sévères de tous les départements, mère de toutes les régions, un amendement qui intervient dans un contexte de baisse drastique des dotations région revient à mettre en place un régime dérogatoire pour la métropole de Lyon alors que tout, que toutes les régions et de toutes les discussions sur les admissions sur les relations avec les collectivités locales le ministre de l'Intérieur avait répété qu'il convenait d'écarter tout pratique d'exception afin de garder une vision d'ensemble, d'où la proposition de suppression. Très bien donc amendement en discussion commune mais en fait ils sont identiques, que monsieur de Montgolfier pour la commission des finances. On a déjà été exprimée donc est-ce que concrètement cette spécificité régionale est liée à transfert de compétences transport manifestement pas, donc on a beaucoup un petit peu de mal à trouver la justification et en tous les cas, c'est en contradiction avec la volonté de renforcer l'échelon régional, en lui attribuant des ressources dynamiques et la est une ressource dynamique, donc évidemment pour ces raisons, vous comprendrez que la commission souhaite comme les présidents amendements supprimé l'article 41 bis qui crée une bizarrerie et qui est en contradiction avec un objectif de donner des ressources dynamiques en région et en plus pas justifiés par transfert d'une compétence. Donc la ligne du gouvernement sur ces amendements identiques mais la Mini. Oui merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les énarques. Comme vous l'imaginez l'avis du gouvernement, est opposé à celui du rapporteur général et donc, considère que la métropole de Lyon comme cause collectivités à statut particulier qui exerce des compétences généralement dévolues aux départements, ainsi que des compétences métropolitaines renforcées justifie la répartition différente spécifique de la CDM donc donc défavorable à l'amendement.

et tout ne doit pas forcément venir de façon identique dans les rapprochements éventuel entre les collectivités, ici les métropole et les départements pourront se faire sur une base volontaire ou doivent pouvoir se faire sur une base volontaire, je note simplement que sauf explication contraire la métropole de Lyon est dans une configuration inédite à ce stade, mais inédite sur le territoire national, il s'agit d'un casse oui generis d'intercommunalité puisque elle exerce à la fois la compèt en même temps, la compétence du département, on ne peut pas plaider sans cesse pour une autonomie croissante dans l'organisation des des territoires et à chaque fois qu'il y a une innovation rétorquer que c'est une rupture d'égalité et et je ne partage pas mais je comprends mais je ne partage pas l'avis de de Monsieur Bocquet, sur l'histoire des 2 vitesses, c'est-à-dire que si à chaque fois il y a des choses un peu différent, qui se passe sur le territoire qu'on expérimente, on dit : avez vous fait alors des des territoires à 2 vitesses, je trouve que ce discours et et contradictoire la métropolisation du pays, c'est qu'il y a des débats là-dessus que ça peut susciter des interrogations nécessite quand même d'en tirer les conséquences en matière d'organisation quand cela est justifié notamment en matière financière et puis en matière aussi administrative c'est donc une adaptation locale qui préfigure aussi qu'une fiscalité, un peu plus souple, un peu plus adapté au territoire pourrait voir le jour, et sans que cela, bien sûr, s'impose à toutes les autres métropoles ou à toutes les autres collectivités pour répondre à votre argument Monsieur rapporteur général, on peut faire du cas par cas, c'était évidemment sous réserve d'évolution éventuelle sur d'autres territoires, mais cela ne nous interdit pas lorsqu'il y a expérimentation lorsqu'il y a un cas particulier d'en tirer les conséquences sur le territoire faute alors ou alors sauf à dire à chaque fois, hé bien on refuse en réalité les expérimentations.

là il y a pas de problème pas expérimenter, mais ce matin, nous défendions l'amendement avec Françoise Hugues a-t-elle sur l'Opinel précisément en demandant une expérimentation, on nous expliquait que c'était pas possible, donc je trouve ça pour le moins étonnant.

monsieur le président je voterai bien sûr cet amendement et je je m'étonne au passage que pour la région Île-de-France, ou les départements qui n'exerçait pas la compétence transports ce sont quand même vu prélever leurs ressources de qu'il l'aurait rétrocédé sur la base 2016 en ayant perdu la dynamique de la de la recette, alors qu'ils avaient bien sûr des recettes des dépenses en pleine dynamique, notamment dans le domaine social, on n'est pas fait non plus d'exception, donc d'exception pour

sur ces amendements identiques. Donc, soutenu par la Commission : avis défavorable du gouvernement qui est pour.

Donc commandement adopté ce qui supprime l'article 41 bis. Alors après, c'est parti, qui n'existe plus. Donc, amendement 674 Madame polluant. Merci Monsieur le Président, la loi notre instituée lors de la création de la métropole du Grand Paris une neutralité financière entre les villes, les établissements publics territoriaux et ladite métropole à cette fin dans la relation entre les établissements publics territoriaux et la NGP une dotation d'équilibre a été créé sur l'ensemble de la métropole du Grand Paris, le montant des dotations d'équilibre et de 924,6 millions d'euros, alors je pas rentrer dans le détail du calcul et qui est présenté dans l'exposé des motifs de de l'amendement, mais je vous dirais qu'un des éléments du calcul de cette dotation d'équilibre est la dotation d'intercommunalité perçues par les anciens du PCI en 2015. Et cette neutralité financière, elle est limitée dans le temps dans l'article 59 de la loi nôtre et notre amendement propose de supprimer cette limite afin d'assurer la continuité des ressources D il est bon de rappeler que les. Philippe financier des établissements publics territoriaux doit être assurée par les villes membres pour assurer la continuité des services publics qui sont portés aujourd'hui et qui doivent l'être demain pour le PT 12 par exemple, qui regroupent 24 villes 3 ex-PCI 700000 habitants, cela représente un montant de 14,8 millions d'euros par an et ça va risquer de déséquilibrer le budget 2018, qui est en cours d'élaboration, il y a, et tout le monde le sait, des annonces qui vont être faites par les de de du mois de janvier pour annoncer une réforme du fonctionnement du périmètre de la métropole du Grand Paris des 2, bref un bouleversement à nouveau institutionnel sur la la, qui toucherait peut-être jusqu'aux frontières de la limite de la région Île-de-France, il nous semble plus raisonnables dans l'attente de ces heures annonce : il nous semble important de ne pas déstabiliser le le déficit l'équilibre qui existe et puis dans la réforme annoncée, il sera temps de revoir les équilibres entre les différentes institutions en fonction de ses quelles seront merci. Oui, sur cet amendement, l'avis de la Commission, monsieur rapporteur général.

est-ce qu'au détour d'un amendement, on peut modifier l'équilibre qui a été trouvé en 2015, n'a pas paru très raisonnable, la Commission, qui est défavorable à cette amendement.

Alors, nous souhaiterions que après. Les l'. Prise de parole forte du président de la République sur la volonté de renforcer le rôle du Parlement en terme de contrôle et d'évaluation qu'on puisse effectivement prendre en compte. Dans le cadre de l'évolution du CICE, hé bien l'évaluation qui a été menée sous l'égide de France Stratégie avec je crois une une constitution de cette commune de ce comité de de suivi. Assez pluraliste, une sélection par appel d'offres de 3 équipes de recherche universitaire indépendant qui a travaillé, qui a posé un certain nombre de conclusions alors quelles sont-elles, le CICR a-t-il permis de redresser notre balance commerciale, la réponse est : nous, les travaux d'évaluation sur les exportations des entreprises déjà exportatrices montres qu'il est, avec un effet quasi nul sur le volume d'exportations des entreprises déjà exportateurs déjà pardon exportatrice, a-t-il permis à des entreprises qui n'exportait pas de s'orienter vers l'exportation, la réponse est aussi négative avec une précision qui devrait être enfin entendus, je cite, la décision d'exporter semblent peu sensibles au coût salarial unitaire, la baisse du coût du travail n'influe pas de façon majeure dans la compétition internationale. Est-ce que le CICE a eu un impact positif sur les salaires et, là aussi, le comité semble indiquer que l'effet positif n'existe que pour les cadres et les professions intellectuelles. Les créations d'emplois espérés se sont-elles réalisées l'estimation des créations d'emplois par ce comité de suivi se situe dans une fourchette de 10 à 200000 emplois sur la période 2013, 2015 le chiffre retenu est de 100000 emplois sauvegardés ou créés sur toute cette période, alors le calcul est facile à faire je vous renvoie à nos récents débats sur les contrats aidés alors Madame la Ministre, pour une fois que nous avons prévu au moment du vote de cette loi, une procédure d'évaluation que tout le monde il faut. le l'évaluation du Parlement puisse être davantage mis en oeuvre, il me semble indispensable d'en tenir compte c'est pourquoi cet amendement, vous propose de retenir donc les conclusions de faire évoluer le CICE en le conditionnant à des 2 pensent qu'ils sont utiles pour l'emploi qui amélioreront la compétitivité de nos entreprises et accentuera l'orientation de notre économie vers une économie plus durable, je vous remercie. Merci. Donc, avis de la commission. vous connaissez la position de la commission des finances, qui n'est absolument pas fanatique du CICE vous savez aussi pourquoi on va dire les choses, le CIC a été mis en place tout simplement pour des raisons budgétaires, il était préférable de prévoir un crédit d'impôt avec et Nene décalage à une réduction de charges, et la preuve, on était obligé d'inventer des dispositifs d'une complexité extrême comme la mobilisation des créances fiscales par la BPI, parce que la majorité sénatoriale, nous partageons l'idée que, il est plus simple d'avoir une baisse de charges ce qui interviendra, c'est à la fois plus lisible, c'est au moins ciblés directement sur le coût du travail il y a pas tous ces problèmes de l'éligibilité de savoir ce qu'on fait du CICE c'était utile en terme de comparaison internationale, puisque quand on regarde le coût du travail chargé,

le coût du travail, les charges et surtout si ces charges sont diminués, donc c'était pour ces raisons n'est évidemment beaucoup plus favorable à la baisse des charges au CICE pour autant, faut-il qu'aurait carrément le supprimer dès 2018, bon évidemment l'amendement du groupe communiste, on ne peut pas et souscrire on nous nous approuvons précisément le basculement du CICE vers la baisse des charges des aides sociales patronales qui permettra de diminuer le coût du travail, d'améliorer la comparaison entre la France et ses voisins et donc avis défavorable sur le 465 l'amendement 595 qui avait présenté à l'instant, il va au contraire complexifier le dispositif, avoir une baisse de charge simple c'est beaucoup plus lisible que d'avoir un CICE conditionnée à l'engagement dépenses relatives à l'innovation et du pays Minergie la formation des salariés, j'ai peur qu'on ait 18 Yves extrêmement complexe qui ne soit pas plus efficace jeu beaucoup plus efficace de diminuer les cherche sociale ce qui ce qui va ce qui va être fait et de transformer le CICE en baisses de charges, c'est ce qui va être fait, plutôt que de vouloir complexifié alors à l'envi le dispositif en lui rajoutant des conditions dont le suivi sera pas forcément évident, donc avis défavorable sur les 595. Merci du gouvernement, même le ministre. Oui merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, du 465. Comme le dit le rapporteur général, la suppression du CICE est déjà une mesure centrale prévue à l'article 40 du du projet doit de finances pour 2018 et conformément à l'engagement du président de la République, ce dispositif serait remplacé par un allégement de cotisations sociales qui sera instauré dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 et permettra d'accroître l'efficacité du soutien accordé aux entreprises, donc nous sommes-nous nous demander, nous Donc, c'est bien évidemment une une une proposition qui qui reste extrêmement complexe. Il ne nous sommes pas abouti, juridiquement, elle introduit une nouvelle assiette pour les dépenses de recherche et l'innovation en laissant subsister la cette constituer des rémunérations versées aux ça varier jusqu'à des véhicules 5 fois le SMIC. Sans se préoccuper de savoir si cela n'aboutirait pas à prendre en compte 2 fois les mêmes dépenses. Donc ça me ça semble complexe et et pas totalement abouti, nous considérons qu'il ne qu'une fusion entre le hier, elle s'est hissée à terme n'est pas approprié. Qu'il faut maintenir des outils différents sur les 2 types d'objectifs : d'une part, l'abaissement du coût du travail pour les entreprises et, d'autre part les incitations aux actions d'innovation et de R&D et donc défavorable également sur le 595. Bien sûr, c'est 2 amendements Madame Lienemann. C'est un débat important parce que c'est le débat sur l'idée qu'on se fait la compétitivité française, c'est notre modèle social, on nous a expliqué quand on est au lancer le CICR, vous savez ça fait débat dans notre assemblée et dans l'opinion que la baisse du coût du travail, j'aime pas ce terme parce que pour moi, je travaille ça dévore une production est plus qu'un coup là cela pseudo baisse enfin la baisse du pseudo, coût du travail allait être un élément déterminant de compétitivité. Force est de constater que telle n'est pas le cas. Les analyses même sur la restauration des marges des entreprises montrent que ça a été à peu près identique dans tous les pays de l'Union européenne et que ça n'est pas liée à ce mécanisme-là puisque d'ailleurs, certaines entreprises ont très peu de salariés ont récupéré beaucoup de marge, donc on est dans un mécanisme où le comité de suivi qui nous était promis comme le moment de faire le rendez-vous sur l'efficacité et plus que circonspect, car non seulement le l'argent mis pour chaque création d'emplois est une ruine mais deuxièmement, globalement, on a, on n'apprend rien gagné sur le terrain industriel qui est un élément déterminant de notre avenir commun, on a toujours plaidé, et je crois que c'est dans la filiation de ce de ce mouvement qu'il fallait conditionner les aides, elle est ciblée ciblées, notamment dans les secteurs menacé par l'exportation, la compétition, la compétition mondiale ciblée vers la réindustrialisation conditionné sur un certain nombre de critères, qui n'était pas d'ailleurs que la création d'emploi parce que la robotisation, la modernisation de l'outil et notre capacité à être plus compétitif est un élément qui, parfois, hélas, va au rebours de l'emploi, mais qui est une façon de prévoir notre avenir. Le gouvernement qui, on a eu ce débat déjà nous explique qu'on va continuer sur la baisse du coût du travail et d'ailleurs, au passage, a refusé des propositions que nous faisions pour soutenir la robotisation, la modernisation de l'outil productif. Alors vous savez, nous on n'est pas plus royaliste que le roi, on préférerait que ça marche. Oui, on est socialiste, oui, moi j'assume pleinement hein. Oui, mais on, on c'est une formule plus royaliste que le roi plus républicain que la République, c'est difficile parce que la République n'est jamais atteinte, mais en tout cas, soyons nous ne sommes pas sectaires sur les méthodes. Simplement, nous constatons que ça finit par fragiliser le modèle social et que ça ne crée pas de compétitivité et de rayonnement économique supplémentaire, donc nous avons essayé de recentrer ce dispositif sur des critères qui permettent de dire, bien sûr, certaines entreprises ont besoin d'être pas toute panne importe comment pas sans ciblage pas sans contrepartie.

Juste 2 mots pour dire que nous maintenons l'amendement et que j'ai beaucoup entendu pendant ces ces débats sur le projet de loi de finances, qu'il y avait une véritable addiction à la dépense publique, moi je crois qu'il y a une véritable addiction à la baisse de cotisations en général comme ça sans sans aucun ciblage et je pense que c'est un vrai problème. Donc merci, c'est pas d'autres explications de vote, je vais mettre, on voit ces 2 amendements de 465 de Monsieur Bocquet donc avec 2 avis défavorables de la Commission et du gouvernement qui est pour. C'est con. Abstention : il n'est pas adopté le 595 fructifier même chose avec 2 avis défavorables du gouvernement de la Commission. Qui est pour.

Alors ensuite le 423 donc Madame remédie. Merci monsieur le président, cet amendement propose de maintenir le taux du CICE à 7 pourcent en 2018 afin de permettre aux entreprises d'amortir le coût de la transformation, en baisse de charges en 2019, d'une part la baisse d'un point du taux de crédit d'impôts en 2018 entraîne pour les entreprises, une perte de 3,1 milliards d'euros d'autre part, la transformation du CICE en baisses de charges pérennes dès 2019 se traduira par une augmentation des prélèvements pesant sur les entreprises, yes participation est forfait social la perte pour les entreprises est estimé entre 5 et 7 milliards d'euros, notamment sur les salaires compris entre 1,5 et 2,5 SMIC pour ces raisons, il convient de maintenir le taux de CICE à son taux actuel.

Oui, il s'agit de maintenir le le comité d'évaluation qui suit les résultats du du CICE pour qu'ils puissent terminer ses ses travaux, ensuite je passe, il faudra le le maintenir jusqu'au bout, mais au moment où ce dispositif se maintiennent maintenons l'évaluation scientifique pour avoir la totalité des, des résultats des études. Donc sur ces amendements, l'avis de la Commission, monsieur de Montgolfier.

le coût de l'amendement serait évidemment assez incompatible déviances publics parce que si on votait cette amendement ça sera dur par à-coups de 3 milliards d'euros supplémentaires pour le budget de l'État, donc on n'a pas ce soir, suffisamment d'imagination pour trouver 3 milliards d'euros d'économies et comme le choix du Sénat, c'est ne pas dégrader le solde donc c'est malheureusement une demande de retrait pour cette raison. L'amendement du groupe communiste, lui, il augmente bien le soldat d'ailleurs Jean-Marc alors là c'est je,

donc je pense que c'est une première, hein, ce soir, donc il est 17 heures 56 le 8 décembre donc, il faut le noter procès-verbal maintenant, le groupe communiste va nous proposer désormais des amendements pour améliorer le solde budgétaire donc d'être noté Madame Lise entendu donc alors on pourrait y souscrire, c'est une bonne idée, mais malheureusement il est la meilleure, sans doute le solde mais il dégrade les comptes des entreprises et donc malheureusement à notre grand regret : avis défavorable, donc, en tout cas je note, c'est évolution et mérite d'être salué, il s'est passé quelque chose, ce 8 décembre à 17

Très bien, Madame la Ministre, l'avis du gouvernement. qui modifie dans des sens contraires, je crois, les taux du CIC, bon ben on va retrouver un bon équilibre est resté sur la proposition du gouvernement, ça me semble plus simple et ça correspond à l'équilibre d'ensemble du dispositif qui a été, qui a fait l'objet de de l'engagement du président de la République s'agissant du du rapport et de le prolonger pour un an, OK, on on évalue un dispositif qui, c'est on va dire sagesse également. Bien, il n'y a pas de prise de parole pour les explications de vote, je vais mettre au pouvoir. Donc l'amendement 423 avec une demande de retrait de la Commission, un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Donc il n'est pas adopté le 462 avec qui avait 2 avis défavorables de la commission du gouvernement qui est pour. pour. Est contre. Il n'est pas adoptée et le dernier le 508 avec 2 avis de sagesse de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Oui, alors attendez on vont saveur réveiller je vous vois pas trop l'intérêt de faire un essai de Bulat suivre quand même le faire. Donc, je vais reprendre, c'est un avis de sagesse de la Commission et du gouvernement qui est pour, debout, s'il vous plaît.

L'article 42 qui est pour. Oui. Oui, qui est contre. Donc, l'article 42 est adopté.

Ces techniques en un mot, il s'agit d'actualiser le régime du nantissement de créances des kinés du crédit d'impôt recherche du CCE et Direct de report en arrière des déficits. L'avis du gouvernement. Merci Monsieur le Président, oui cette mesure permet de continuer à inciter les banques à acquérir ces créances fiscales, faute de pouvoir aujourd'hui se refinancer auprès de la Banque de France, avec ces créances, elles y renoncent parfois donc favorable.

43. Ces contrats. Donc, l'article 43 est adoptée après l'article 43 bis. Un amendement du gouvernement le 715 Madame la ministre. donc c'est c'est un amendement de coordination qui allège la rédaction d'Arte, l'article 231 du CGI sans modifier son sens. Monsieur monde avis favorable. Donc je je vais auparavant demandé Madame la ministre sur le vote précédent il est-ce que vous levez le gage, puisque vous étiez favorable à l'amendement de la commission de Monsieur Montgolfier donc je suppose que oui merci, donc, sur cet amendement, qui est celui du gouvernement le 715 il n'y a pas de l'explication de vote donc avec un avis favorable de la commission jamais aux voix qui est pour. Les comptes. Il est adopté. Alors on va voter l'article 43 bis qui est donc légèrement modifié et qui est, pour l'article 43 bis. Qui Ci-contre. Donc il est adopté. L'article 43 ter un amendement du gouvernement le 714 semaines le Ministre. Oui, Monsieur le Président, à nouveau, un amendement de de coordination qui corrige la rédaction initiale de l'article 43 terre pour modifier dans le sujet d'article 1679. Favorable. Donc, qu'est-ce qu'il y a des explications oui Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président sur sur cet amendement 714 je voudrais exprimer l'opposition notre. Ce groupe qui suit, Valérie Létard sur ce dossier car cet amendement finalement supprime le ITS au dépend des responsables privés non lucratifs du Champ sanitaire, sociale et médico-sociale, donc, il semblerait que, au lieu d'une dinde un rédactionnel ou d'un amendement assez simple : en réalité, cet amendement affecte affecte cette disposition de façon trop importante, donc notre groupe qui est opposé, suivant le souhait notamment du chef de file en la matière qui Valérie Létard. Oui, madame propecia. Même même position puisque, selon les informations que l'on reçoit ça aurait des incidences mais au moins 50 Madame la Ministre souhaitez répondent. Je confirme qu'il s'agit de pure pur coordination pour cet amendement. Monsieur. Monsieur de Montgolfier. Pour bien préciser les choses, je sais qu'il y a eu un certain nombre de collègues ont reçu des interventions de l'UDS peine il serait pénaliserait les établissements médico-sociaux, les exclure du bénéfice du CTS et en tous les cas, on a bien regardé les choses, la commission des finances de la la regarder et je peux vous confirmer que ce n'est pas notre papa tation le grondement vient de confirmer la pure coordination

y a pas d'autre explication de vote, donc je vais mettre aux voix cet amendement qui a un avis favorable de la commission. Et pour. Ces contrats. Donc il est adopté. Et l'article donc prend la rédaction effectivement. De l'amendement.

entre la Commission européenne et la Grande-Bretagne sur les modalités concrètes du Brexit progresse, bon un divorce n'est n'est jamais heureuse mais il on nous n'avons pas intérêt à ce qui se passe le plus mal possible, en revanche, il a une conséquence, c'est qu'il rebat les cartes entre les places financières du continent européen et la récente annonce de la localisation de l'agence bancaire européenne à Paris est une excellente nouvelle dont nous nous félicitons tous je pense, l'attractivité de la place de Paris était déjà présent en première partie de notre PLF, vous vous en souvenez, avec l'article 15 où nous avons supprimé l'extension de de la taxe sur les transactions financières aux transactions infra-journalières pour des raisons à la fois techniques et également de signal économique alors cet article 44 ne concerne pas les produits cette fois mais les talents puisqu'il consiste à supprimer la surtaxe de 20 pourcent du barème de la taxe sur les salaires appliquée et de revenir au taux de 13,6 au-delà des seuils, l'enjeu est d'attirer les cadres supérieurs à Paris et en Île-de-France ces prochains mois et ces prochaines années car le Brexit prendra du temps, nous, nous le savons, une récente étude du Conseil d'analyse économique, cherche à évaluer la place de Paris dans la concurrence européenne Paris constitue une place financière, de taille semblable à Francfort mais nous attirons nettement moins de filiales de groupes étrangers en comparaison à d'autres centres financiers européens si le vivier des compétences et des emplois qualifiés et très important en Île-de-France, c'est un atout pour l'Île-de-France, nous sommes pénalisés par l'accès perfectible entre les aéroports et Paris et aussi une partie de notre fiscalité et du coût du travail, s'agissant de la fiscalité et je reviens donc à l'article 44 l'taxe sur la salaire est un substitut à la TVA, pour le secteur financier, puisque celui-ci en est exonéré mais nous pourrions-nous demander demain et après d'ailleurs des évaluations pour savoir si c'est un bon substitut parce que la prod la progressivité de la taxe sur les salaires est-elle encore pertinente au regard de la TVA qu'elle remplace et qui est-elle proportionnelle comme vous le savez, la piste d'une simplification sur la taxe sur les salaires avec un taux peut-être unique mériterait d'être étudiée donc vous l'aurez compris le groupe la République en marche, soutient l'article 44. Le 463 Monsieur Bocquet. Mais il ne se privant, vous l'aurez compris le groupe CRC ne soutient pas cette partie 44, ça n'est une surprise pour personne parce que là on parle quand même de la suppression du taux supérieur de la taxe sur les salaires alors que rappelons les chiffre quand même, je crois qu'on est au-delà des 12689 euros mensuels, le salaire médian 1600 euros en France à peu près, je connais des gens à 1600 euros extrêmement talentueux dans leur discipline, voilà donc je vois bien que ça fait partie du paquet compétitivité attractivité de la place financière de Paris dans la grande compétition ouverte après la fuite des banquiers de la City, c'est pas fait à mon avis, c'est pas fait, voilà donc les gros salaires Nasri financière viendrait donc ça stagne à Paris, notamment parce qu'il faut de l'argent pour se payer les talents, c'est une logique on ne partage pas du tout, et donc on propose la suppression thématique 44 pour ces raisons-là.

parce que cette suppression s'inscrit effectivement dans cette volonté d'être attractif de concurrencer les Britanniques pour récupérer les les entreprises, la City Mais est-ce que vous pensez vraiment que ça va pouvoir se faire sur la base de cette la suppression de cette taxe sur les salaires de plus de 150 2200 119 euros annuels. Est-ce que le Royaume-Uni va rester sans réaction, mais non, le gouvernement britannique a déjà annoncé des mesures d'allégements fiscaux, encore plus importante alors cette idéologie du moins-disant fiscal et social va nous amener toujours plus loin, toujours plus loin vers des étapes supplémentaires de réduction des taxes, des impôts et cotisations alors d'un côté on dit il faut lutter contre le dumping social et fiscal que nous constatons en Europe et puis d'un autre côté, on le fait, vous participez à cette course au moins disant fiscal mais nous pensons que la qualité de la formation de nos ingénieurs, nos experts financiers de nos infrastructures sont les garants de l'attractivité de la France, donc il faut marquer un coup d'arrêt à cette politique parce que ça nous mènera, c'est sur un déséquilibre de notre système de protection sociale à moins que ce ne soit ce qu'on souhaite. bon, vous connaissez la la la vie la Commission puisque ceux qui sont à laquelle qualifiant des finances n'ont participé à la restitution des travaux du groupe de travail que nous avions mené sur la fiscalité et la surtout la compétitivité de la place de Paris postérieur au Brexit, c'est un travail qui a été menée qui a été menée collectivement et moi j'ai pas beaucoup participé en signant un rapport et qui ce qu'il ressort une partie de ce qu'a dit Julien Bargeton c'est-à-dire, concrètement, nous avons un vrai problème de comparaison par rapport à Francfort, il se joue bien sûr sur la seule sur la fiscalité, il se joue sur les différentiels de charges sociales,

il se joue tout sur notre image d'instabilité fiscale et malheureusement, quand j'ai été amené, dans ce cas de ce travail, a rencontré des dizaines et des dizaines et dizaines d'acteurs en France et en Europe aussi bien qu'en Asie et 10 : toujours le problème en France c'est que vous êtes amené à changer et à modifier en permanence votre fils qui a été parfois de trajectoire, alors là il y a une trajectoire sur la baisse de l'impôt sur les sociétés, il faut maintenir, il y a d'autres trajectoire qui sont abaissées mais avant tout ce qu'il faut offrir un cadre stable face à des pays qui, comme l'Irlande font de leurs taux bas de fiscalité,

les payé par les entreprises qui, comme vous l'avez dit, ne payent pas la, la, la TVA et dans la dernière tranche la tranche la plus élevée, c'est à 80 pourcent à peu près la l'industrie financière, la seule différence, c'est que si vous avez très concrètement à salaire d'assez d'un cadre de haut niveau

et évidemment Paris en plus cette action et salaires hé bien évidemment c'est une, c'est un élément de compétitivité qui font que les annonces de délocalisation qui interviendront pour partie nécessairement accapare du passeport se font plus vers l'Allemagne notamment ouvert des pays il n'y a pas de fonction et salaire donc cette mesure, je l'avais préconisées dans le rapport, le le garnement la retenue avec d'autres, je, je, je pense que c'est un élément essentiel du débat et revenir dessus, ce serait totalement contreproductif à un moment où les décisions vont se prendre parce que autre jour nous entendions Michel Barnier vous le rappeler la date malheureusement du divorce avec le Blatter et devait inéluctable et avec la part du père sport ça obligera à délocaliser

attendu un élément qui sera visible, un élément qui arrive au moment où les décisions des banques se prennent, nous avons une pente à remonter à l'égard de et de d'autres villes

publication de vote pour moi il n'y a pas d'ambiguïté : je suis évidemment pour la défense de l'attractivité de Paris, je considère que ce serait une mauvaise mesure mais je voudrais avoir simplement une explication putain c'est tout simplement de cohérence à l'issue des élections sénatoriales qui viennent de se tenir à Paris parce que nous sommes un certain nombres d'élus parisiens dans cet hémicycle, on a une vision plus ou moins différente de l'attractivité, mais j'ai cru comprendre que Madame Hidalgo au nom de l'attractivité défendait le principe de la suppression de cette taxe, en tant que maire de Paris, lorsqu'elle est à côté du 1er ministre et parallèlement la liste qu'elle soutient, 2 des 4 membres de la liste sont contre cette attitude de madame la maire de Paris alors j'aimerais que moi naïvement étant un élu je dirais de l'opposition municipale, même si c'est la majorité sénatoriale qu'on m'éclaire un petit peu parce que je n'y comprends plus rien, je voudrais bien savoir si la municipalité parisienne est favorable à la suppression de cette taxe, comme semblent le dire Madame le maire de Paris, ou si au contraire, les élus socialistes parisiens, soutenus par Madame Hidalgo sont défavorables à cette taxe, j'aimerai bien vraiment que quelqu'un puisse m'éclairer à l'occasion de ce débat parce que je reconnais que le double langage par moment ça agace. Merci donc, explications de vote Madame Goulet. j'ai eu à rencontrer les agences de notation et les agences de notation, qui nous ont dégradé, il y a quelques années, 2, 3 et qui nous ont désormais dégradé ont une un examen extrêmement attentif de votre politique fiscale, ils ont aussi un examen extrêmement attentif de la façon dont on gère notre fiscalité, de façon totalement erratique. En étant absolument incapable d'avoir une visibilité à plus d'un PLF ou d'un PLFR et donc je pense que de ce point de vue-là la stabilité fiscale est une est est vraiment un élément d'attractivité du territoire qu'qui soient bon mauvais après on peut, on peut en discuter, pas avoir le même avis sur des dispositions, mais on ne peut pas prétendre à une attractivité du territoire en modifiant systématiquement les règles du jeu. ça, c'est complètement impossible et et les agences de notation nous scrute c'est pas Big Brothers, mais ça finit par y ressembler je pense, comme l'a dit le rapporteur général que cette que cette stabilité fiscale est vraiment un élément fondamental de l'attractivité donc suivre évidemment la commission sur ces amendements. Très bien, il n'y a pas d'autre explication de de vote. Sur ces 2 amendements, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRCE sur les amendements 463 et 664.

Le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter, donc le scrutin est clos et j'invite les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

y a aussi les résultats du scrutin numéro 40 sur les amendements identiques 463 664 conclut l'ensemble délégation de vote accordé par les sénateurs vont politique et notifié la présidence nombre de votants 340 suffrages exprimés, 335 pour l'adoption 88 contre 247 donc, que le Sénat n'a pas adopter ces amendements. Nous avons ensuite 4 amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune le 507 monsieur Oui merci monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, puis si votre accord peut-être il y a 2 amendements qui se suivent, je peux puisque sans continuité. un peu les présenter dans le même ordre d'idées pour modifier le code général et des impôts, et ce sont des amendements, contrairement au précédent, donc pour maintenir néanmoins l'article 44 liée à la taxe sur sur les salaires et puis naturellement pour favoriser l'implantation en France, le cadres étrangers à fort potentiel, par mesure d'équité, de proposer de relever le plafond de la tranche médiane est de créer une franchise dans le cadre de la taxe sur les salaires, on ne la rendant applicable que pour la France, fraction des salaires excédant 7721 euros, soit le seuil actuel d'application du tout, moi j'aurais de 8,5 pourcent puis également dans un souci de neutralité budgétaire cet amendement propose. De rehausser le taux de la tranche le plus haute à due concurrence de la baisse des recettes publiques provoquée par cet amendement, qui propose également que la baisse de taxation proposée par le gouvernement soient davantage ciblées sur les salaires médians sont et l'objectif de l'article 44 le suivant la l'amendement 482 rectifier donc aussi à l'initiative de notre collègue monsieur on perd et plusieurs d'entre nous, également, c'est aussi pour proposer naturellement dans la continuité de rehausser le taux de la tranche également pour compenser la diminution de recettes due à la suppression de la première tranche qui qu'introduit l'amendement et qui permet aussi une simplification de la rédaction des articles concernés du code

Oui, monsieur le président, mes chers collègues, il a été fort bien défendu par notre confrère Marc Laménie, vous avez très bien compris le sens de cet amendement, j'en profite, juste pour vous rappeler qu'effectivement les indépendants sont tout à fait favorable à l'article 44 et au mécanisme qui introduit, qui va permettre une attractivité de notre territoire et contrairement à ce qui a pu être pensé par certains qui va amener plus de ressources sur notre territoire, puisque l'objectif c'est d'attirer des nouveaux salariés et donc d'attirer de nouvelles ressources et donc pour notre système de sécurité sociale d'attirer plus de cotisations, c'est ça l'objectif, au final, la France et l'ensemble des Français y sont donc gagnants du reste, je ne crois pas que les Allemands qui sont plus compétitifs sur par rapport à nous sur les salaires, soit dans une situation calamiteuse ou inquiétantes quant à la protection sociale de leurs salariés, donc de tenter de rattraper une toute petite partie du retard que nous avons sur eux en terme d'attractivité fiscale, ça c'est l'objectif de l'article 44 que nous partageons totalement l'amendement qui vous est proposé introduit juste en complément je dirai même, et le terme est parfaitement adéquat dans le même temps une équité fiscale en proposant une franchise sur les salaires les plus modestes, donc on toucherait donc aux salaires les plus élevées et une franchise de taxe sur les salaires les plus modestes, afin d'équilibrer l'ensemble, voilà l'esprit de cet

complément et en rappelant que dans un souci de neutralité budgétaire, c'est aussi une volonté de tempérer la diminution du taux de la tranche la plus haute tranche supérieure à 150 2279 euros pour compenser la diminution de recettes due à la suppression de la première tranche qu'introduit l'amendement et aussi dans un souci de simplification jour merci. Merci donc l'avis de la Commission sur ces quatre s'amendement de bombes identique Monsieur Montgolfier. ces amendements proposent c'est tout à fait sympathique en soi de supprimer, non pas la dernière tranche, mais la 1ère tranche de la taxe sur les salaires mais pour compenser le cours de m'édifier le barème de cette action, les salaires bonsoir évidemment des uns fait induit puisque concrètement relevant en modifiant le le la dernière tranche : ce serait défavorable aux plus hauts salaires, donc ce serait des effets induits je remarque, on a tout à l'heure parler de de la baisse de charges versus CICE dans les arguments qui sont en faveur de, de, de la baisse des charges, il y a évidemment le fait que la baisse des charges va concerner le monde associatif qui n'étaient pas concernés par le CICE, donc, et qui va bénéficier de la baisse de charges, donc c'est une mesure supplémentaire, donc je ne veux pas à mon sens, modifier l'actuel barème n'ayant ce qu'on a dit tout à l'heure sur la tranche la plus élevée, qui concernait essentiellement à 80 pourcent l'industrie financière, et donc c'est de de retrait sur ces amendements. Madame la ministre, l'avis du gouvernement.

les autres salaires qui supporteront donc des taux majoré de façon très significative sur ce qui va bien sûr à l'encontre de l'objectif poursuivi par le gouvernement en supprimant la la 4ème tranche donc avis du défavorable du gouvernement sur sur ces amendements. ces, sur ces amendements est-ce que je mets aux voix est-ce qu'il y a des retraits. et puis c'est aussi un comme on dit, on est en vie en loi de finances en regardant aussi les contraintes financières et je crois que c'est, c'est aussi l'objectif de de de tous et puis vu des explications fournies par notre rapporteur général et de Madame Lamy je retire les 3 amendements.

Oui, simplement pour proposer d'aller jusqu'au 44 sexy assis à 4 amendements, je pense qu'on peut les faire et puis on arrêtera après. Voilà, c'est parfait, 4 amendements, ça peut durer parfois très longtemps et ça peut être très court mais enfin je pense que là, on sera dans l'raisonnables. donc sur l'article additionnel après l'article 44 533. Monsieur de Montgolfier au nom de la commission des finances. Monsieur le rapporteur général au nom de la commission des finances. et malheureusement, vous le savez l'attaque sur les faux salaire constitue reviendra parler à l'instant une spécificité française, il y a pas d'équivalent en Europe, semble-t-il, sauf au Danemark et on vient à l'instant de voter l'article 44 qui constitue un excellent signal sur la dernière tranche, mais une évidemment l'idéal eut été de supprimer totalement la taxe sur les salaires, malheureusement ça coûterait beaucoup trop cher grand regret, c'est 13 milliards 7 d'euros et c'est la raison pour laquelle le rapport que je citais tout à l'heure, propose une mesure forte mais qui serait ciblé sur les impatriés et donc c'est c'est la mesure qui est proposée, études Artic 533 restreinte aux impatriés qui permettrait de ramener à Paris des salariés venant post-Brexit donc c'est une mesure extrêmement favorable à coup évidemment beaucoup beaucoup beaucoup plus limité et conditions ciblage que la suppression totale de la taxe sur les salaires, donc je pense que vraiment vous très favorable n'est-ce pas. Très bien, donc on va voir ça tout de suite l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Merci monsieur le président, monsieur le rapporteur général, malheureusement je ne peux soutenir votre amendement, je partage votre préoccupation quant on avait attractivité de la place financière de Paris, ça a été dit et le gouvernement a déjà fait des choix forts qui vont dans ce sens, en revanche, la mise en place d'une telle mesure de, de, de suppression de la taxe sur les salaires, l'exonération des avec pour les impatriés présentent un risque d'inconstitutionnalité pensent qu'elle constituerait une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les redevables de la taxe sur les salaires. Donc, avis défavorable. Donc sur cet amendement, présenté par la Commission, pas d'explication de vote, donc je vais le métro voit avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour.

Oui, Monsieur le Président, depuis 2 mois que je suis président de notre commission des finances, je regarde de l'intérieur comme d'abord la loi de finance je participerai bien sûr au débat engagé par le gouvernement, et nos collègues députés sur la procédure budgétaire, mais ce sont les conditions d'élaboration de la loi fiscale qui me frappe le plus, nous examinons de manière simultanée des réformes à la fois importante politiquement et lourde techniquement dans un calendrier qui ne permet pas de consultation approfondie et en nous reposant entièrement sur les données chiffrées fournies par le gouvernement, or le gouvernement et son administration même pris dans la machine infernale de la session budgétaire ne sont pas toujours en mesure de nous fournir les données dont nous pensons avoir besoin, quand tu nous en avons besoin, c'est pourquoi je pense qu'il faut ouvrir l'accès aux données et permettre aux parlementaires, mais aussi à tous les acteurs de la vie économique et sociale aux universitaires et chercheurs la possibilité de traiter eux- mêmes les données de faire leurs propres simulations de mesurer l'incidence de la modification de telle ou telle paramètres d'une réforme fiscale, le Sénat a adopté dans la récente loi de programmation des finances publiques, mais un amendement visant à disposer de certaines données dans des formats exploitables, aujourd'hui il s'agit d'aller plus loin et de demander au gouvernement de fournir à l'appui de toutes les réformes fiscales qu'il propose les codes sources traduisant en langage informatique, chacune des dispositions proposées, cela permettrait, je l'ai dit de nourrir le débat public et d'élaborer la loi fiscale de manière plus transparente et éclairé, cela contribuerait aussi à clarifier ce que le gouvernement propose au législateur de voter car le langage informatique permet de lever des ambiguïtés parfois permise par les rédactions littéraire, ce que je dis n'est pas théorique puisque certaines structures aujourd'hui investi dans le codage informatique de la législation de cette manière, réussi à identifier des vice dans la conception de certains dispositifs, ce que je propose serait profondément novateur, révolutionnaire, même au sens où nous traversons une révolution numérique, dans la mesure où la France serait sur ce sujet le 1er pays au monde à aller aussi loin, mais c'est aussi une manière de prendre les devants plutôt que de courir derrière l'évolution de la société, je vous rappelle que, désormais, et en particulier depuis la loi pour une République numérique d'octobre 2016 les codes sources font partie des documents administratifs qui doivent être communiquées sur demande des concitoyens l'algorithme administration poste Bach qui a beaucoup défrayé la chronique, a ainsi dû être rendues publiques ou encore la DG Philippe a dû rendre public le code source de l'impôt sur le revenu, l'administration fiscale française a toujours été exemplaire en matière de numérique et de dématérialisation, faisons en sorte de conserver notre longueur d'avance. et blessé, merci l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur général. Il était évidemment favorable parce que ça va améliorer la formation du Parlement, ça va l'aider à partir de commission des finances, dires des simulations fiables, comme l'a dit le président, ce n'est jamais que l'application Madame la Ministre de la loi de l'article L. 302 du côté des relations entre le public à Nice rations qui prévoit que sont considérés comme de documents administratifs communicables les codes sources donc, dès lors, on ne peut pas le le refuser, mais le mettre en annexe, ce serait évidemment un progrès important et il est bien prévu au type de c'est l'article suivant de l'article plutôt elle 300 tiré 4 que toute mise à disposition, vrai dans un standard ouvert aisément rectifier Abidi zappe, donc c'est ce que nous demandons et je souscris pleinement l'intention du prix, la commission des finances de disposer de ces Ksours, ce serait vraiment une première et en tous les cas une amélioration considérable de la formation du Parlement et de cela d'eau simulation dont nous avons besoin pour voter des lois fiscales fiables. Madame la ministre, l'avis du gouvernement. Si mesdames et messieurs les sénateurs, le gouvernement est défavorable à cet amendement, alors alors pour ce qui concerne la législation fiscale en vigueur ses codes sources sont au moins en théorie, déjà disponible dès lors que depuis la loi pour une République numérique le code-source fait partie des documents administratifs communicables pour les mesures nouvelles et les propositions de loi de finances, la proposition est malheureusement irréaliste dès lors que le code informatique et mis au point en aval de l'adoption de la loi et pour tenir compte des dispositions effectivement adopté on peut c'est c'est c'est une proposition qui nous semble impossible à mettre en oeuvre, à titre d'exemple, l'application de gestion des relations avec les usagers de la fiscalité professionnelle compte environ 4 millions de lignes de code et une modification législative peut nécessiter sa modification dans quelques milliers de programmes unitaire. Donc on a besoin de ce temps technique après l'adoption de la loi pour mettre en oeuvre dans les codes informatiques et donc pouvoir être en mesure de les communiquer donc défavorable. Donc sur cet amendement, oui monsieur blessé. Je suis assez surpris de la réponse du gouvernement parce que ce serait une modernisation considérable de nos méthodes de travail moindre une moindre charge pour les services de Bercy qui aujourd'hui sont tenus de nous répondent de façon incessante, si on ne veut pas qu'on le mette dans la loi, moi, je n'hésiterais pas à les demander au type des pouvoirs particuliers, président de la commission et de toute façon, il faudra nous les donner parce qu'aujourd'hui, Madame la Ministre, nous dit qu'ils sont en principe communicable mais son en principe vaut un certain nombre de contentieux au Conseil d'État pour les obtenir, c'est quand même assez particulier comme mise à disposition. Merci, explications de vote Madame Goulet. parce qu'on est aujourd'hui en plus dans une dans une politique générale d'Open Data en plus, on en a besoin pour pour travailler au quotidien et j'ajoute que sur la loi sur la République numérique il y a en plus une brochette de décrets d'application qui sont pas encore sortis, ça tout ça nécessite quand même que le Sénat donne un signal fort et je pense que la meilleure façon de donner un signal, c'est de voter cet amendement 682. Pas d'autres pays, explications de vote, donc je vais mettre aux voix cet amendement avec un avis favorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement donc sur le site 182 qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Donc il est adopté.

il est adopté le 44 terre qui n'a pas été modifiée qui est pour. Abstentions : il est adopté le 44 quater donc nouveau qui est pour. Bon. Abstention donc il est adopté et nous abordons les 2 derniers amendements sur le. 44 qui inquiète alors amendement 534 présenté par Monsieur de Mongolfier au nom de la commission des finances, monsieur le rapporteur général. Amendement vise à maintenir un petit crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale, le coup est limité mais ça ne paraît surtout un très très mauvais signal monsieur Barre, Bargeton à l'égard des PME qui exportent parce que quel est le problème de la France, vous savez très bien, c'est son problème d'exportation, c'est pas les grandes entreprises qui vont bénéficier de ça sont les PME, notamment sa finance. Evie VIE donc c'est très beau et ça aide à l'exportation, notamment des entreprises, c'est un outil utile pour les PME, donc c'est la raison pour laquelle nous souhaitons le maintien du 2 de ces dispositifs de de crédit impôt pour dépenses de prospection commerciale. Merci donc l'avis du gouvernement. Le gouvernement est défavorable à cet amendement, nous souhaitons supprimer ce ce crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale qui n'a pas démontré sa réelle efficacité très positif, très peu utilisé 1600 bénéficiaires relevés par la Cour des contres, dans son rapport public de 2011 pour son caractère redondant avec d'autres aides, voilà, donc nous sommes défavorables à l'amendement. Donc sur cet amendement est-ce qu'il y a des explications de vote, sinon je vais le mettre au pouvoir. Donc un amendement de la commission avec un avis défavorable du gouvernement. Qui est.

Qui s'abstient donc l'amendement est adopté, donc l'article 44 inquiet ce nouveau qui est pour.

C'est pas sujet majeur mais il nous semble que les informations qui sont demandées qui heurta 44 sexy se relève du plus du Cerfa si vous l'exactement les précisions, c'est le numéro 11000 qui empêche les entreprises qui va bénéficier du CIR et on n'a pas, mais dans le code général des impôts, ce type de disposition donc c'est la raison pour laquelle la Commission dans un souci de de rigueur, considère qu'il n'y a pas besoin de mettre dans le CGI des discussions qui n'en relève pas. y a l'avis du gouvernement. les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses de recherche doivent déjà communiquer un certain nombre d'informations sur la nature de leurs travaux pour bénéficier du C. hier et il ne nous sommes pas absurde que cette information est et pas non plus très très lourd que cette information supplémentaire soit fourni ce qui permet, voilà de joindre toute l'information pertinente dans une même déclaration donc défavorable. Pas d'explication de vote sur cet amendement donc amendement de la commission avec un un avis défavorable s'il n'y a pas retrait il est maintenu, monsieur, oui il est maintenu, donc je vois qui est pour cet amendement.

Donc, nous avons joué lever la séance, nous avons examiné 176 amendements cours la journée dans récent 23 à examiner sur ce texte. L'ordre du jour du lundi 11 décembre 2017 à 10 heures 14 heures 30 et le soir suite donc du projet de loi de finances pour 2018 suite de l'examen des articles de la seconde partie non rattachés au crédit, la séance est levée.